La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 25 mars 2021 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation

chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés est parvenue à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République

Monsieur le président du Sénat, monsieur le président de la commission des lois, mesdames les rapporteures, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le ministre de l'éducation nationale, monsieur le garde des sceaux, madame la ministre déléguée, la République est attaquée depuis de nombreuses années par des tenants, ceux du séparatisme, ceux de la radicalisation qui mène au terrorisme. Trois gouvernements successifs, singulièrement des gouvernements qui ont agi à la suite d'attentats meurtriers sur le territoire national, ont pris des dispositions très importantes, législatives et réglementaires, en termes de moyens, pour lutter contre la radicalisation et contre le terrorisme.

le communautarisme, la séparation avec les valeurs et les buts de la République, la radicalisation et le terrorisme, il n'y avait pas de différence de nature. de nature. Nous constatons, et l'odieux assassinat de Samuel Paty est là pour en témoigner, qu'il n'y avait en fait qu'une différence de degré. Dans son discours des Mureaux, le Président de la République a eu l'occasion d'évoquer l'ensemble de l'arsenal législatif et réglementaire regroupant que le gouvernement de la République doit mettre en place, sous son autorité, pour lutter contre ces séparatismes. Si je devais les caricaturer, je dirais que ceux-ci sont de deux ordres, parfois complémentaires, souvent différents.

à tous les services publics : ceux de l'État, qui doivent évidemment en tirer les conséquences, tout comme ceux des collectivités locales. En effet, nous avons tous collectivement à connaître d'un champ de délégation de service public,

nous ne devons toucher les grandes lois et les grands principes de notre État de droit- la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté de culte -qu'avec une main tremblante, mais tout de même assurée, afin de garder l'ordre public. Tel est l'équilibre que nous devons trouver ensemble, mesdames, messieurs les sénateurs, après le travail riche effectué à l'Assemblée nationale. C'est dans cet esprit de compromis républicain et de fermeté républicaine que le Gouvernement se présente à vous.

Nos compatriotes musulmans doivent faire, comme les protestants et les juifs avant eux, une migration vers la loi de 1905, laquelle a ses compromis, ses avantages mais aussi ses inconvénients.

Nous avons bien conscience, mesdames, messieurs les sénateurs, qu'il s'agit d'un texte difficile. En effet, la passion ne manque pas de se déclencher lorsque le législateur touche à l'intime, aux convictions, à la religion, au fait de croire ou de ne pas croire.

Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde nous rappelle la loi de 1905, à commencer par les associations cultuelles. Nous saluons évidemment cet attachement quasi unanime de la République à ce texte. Il ne nous a cependant pas semblé qu'en 1905 tous les cultes étaient très favorables à la loi portée par Aristide Briand

il faut savoir écouter ce qui manque dans la République. Lorsque des personnes qui sont à la tête de structures cultuelles affirment que les juifs sont des mécréants,

les partis politiques, les représentants des cultes, les intellectuels, les associations philosophiques. Il a été examiné par l'Assemblée nationale, qui y a apporté de nombreuses améliorations, après plus de 80 heures de débat dans l'hémicycle et quelque 2 700 amendements. Nous avons eu, depuis lors, des échanges francs avec Mmes les rapporteures, dont je voudrais ici saluer le travail et l'engagement. Nous nous présentons aujourd'hui devant vous avec la même disposition d'esprit et un objectif clair : défendre nos valeurs et la promesse républicaine de laïcité, promesse de liberté, d'émancipation et de progrès, donner à la République les moyens de lutter plus efficacement contre ce que le Président de la République appelle « le terreau du terrorisme ». Nous rappelons ainsi la souveraineté absolue des principes de la République sur tout autre système. Cela passe, bien sûr, par la neutralité des services publics et par un meilleur accompagnement des activités associatives, pour empêcher qu'y prospèrent des discours et des pratiques contraires aux valeurs de la République. Notre mot d'ordre est clair pas un euro d'argent public pour les ennemis de la République. En ce sens, comme l'a voulu le Président de la République, nous proposons la création d'un contrat d'engagement républicain, évoqué par le ministre de l'intérieur à l'instant. Le principe en en est simple : les associations qui souhaitent recevoir une subvention publique s'engageront, par ce texte, à respecter les valeurs de la République ; en cas de non-respect de l'engagement, la subvention pourra être reprise. Ce contrat d'engagement républicain, élaboré avec les élus et les associations, est un contrat de confiance avec le monde associatif. L'immense majorité des associations participent de l'offre républicaine, mais une minorité d'entre elles véhiculent des valeurs contraires aux principes sur lesquels repose la République. Grâce à ce contrat d'engagement républicain, l'État l'État et les collectivités auront à leur main un outil juridique clair. Le respect des principes de la République implique, bien sûr, celui des droits des personnes, et notamment l'égalité entre les femmes et les hommes. Les idéologies séparatistes s'attaquent d'abord aux femmes, en voulant décider à leur place ce qu'elles ont le droit de faire ou de ne pas faire. Ces idéologies ne supportent pas leur liberté, qui préfigure celle de la société dans son ensemble. Nous pensons que toutes les femmes qui vivent en France doivent être respectées dans leur intégrité. Elles doivent toutes être protégées dans leur dignité, dans leur liberté. Le féminisme, c'est de ne pas accepter pour les autres femmes ce que l'on ne tolérerait jamais pour nous-mêmes,

Il y a des années de cela, la France a eu le courage de dire non à l'excision en prenant une loi forte, en montrant la voie à de nombreux pays du monde et en portant ce travail de conviction, la diplomatie féministe. Nous devons aujourd'hui poursuivre ce combat et oser affirmer que la République ne tolère aucune atteinte à la dignité humaine et qu'aucune atteinte à la dignité des femmes n'est excusable au motif de la coutume ou de la pratique. C'est ce que nous vous proposons avec le chapitre III, que l'Assemblée nationale a souhaité intituler « Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l'égalité entre les femmes et les hommes ». Dans ce chapitre, nous veillons à l'égalité de traitement entre héritiers, afin que les filles ne puissent pas être déshéritées. Je tiens à remercier le garde des sceaux pour son engagement personnel sur cette mesure. Nous instaurons également une réserve générale de polygamie pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Nous affirmons que les hommes de nationalité étrangère qui sont coupables de faits de polygamie n'ont rien à faire sur le sol français. Nous voulons également interdire aux professionnels de santé d'établir des certificats de virginité. Les professionnels qui en délivreront seront passibles de poursuites. Je veux être très claire, ce n'est pas en produisant des certificats de virginité, de certificats dits « de complaisance », que nous améliorerons la condition des jeunes femmes victimes de pressions séparatistes. Ce n'est pas en agissant ainsi que nous les protégerons. La commission des lois a d'ailleurs souhaité apporter plusieurs modifications au texte, dans le prolongement des débats de l'Assemblée nationale, pour poursuivre également les personnes qui incitent ou contraignent à cette pratique. Je crois que ces modifications vont dans le bon sens.

Toutes ces dispositions s'accompagneront de politiques publiques fortes pour les concrétiser. Nous y travaillons déjà. Enfin, le ministre de l'intérieur et moi-même avons déposé à l'Assemblée nationale des amendements pour mieux renforcer la laïcité dans le service public.

monsieur le président de la commission des lois, monsieur le président de la commission de la culture, mesdames les rapporteures,

porte une ambition : défendre et protéger notre République contre le fléau du séparatisme, notamment islamiste. Cette ambition pour conforter le respect des principes républicains s'inscrit dans une approche globale portée par chacun de nos ministères : garantir, d'abord, la transmission de ces principes par l'enseignement à l'école prévenir, ensuite, les infractions qui seraient faites à ces principes ; donner, enfin, les moyens juridiques d'une réponse pénale rapide, systématique et adaptée à ces actes qui sapent les principes que nous défendons tous et qui fondent la République française. Ce résultat ne pourra être atteint sans une mobilisation totale de la justice de notre pays. C'est pourquoi je porte au nom de la Chancellerie plusieurs dispositions, qui ont d'ailleurs été maintenues ou enrichies par votre commission des lois. Ainsi, l'article 3 du projet de loi élargit le dispositif du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (Fijait), en y intégrant désormais les infractions d'apologie et de provocation au terrorisme. Il est essentiel, pour renforcer la lutte contre le terrorisme, que toute personne postulant à un emploi ou effectuant une demande d'habilitation fasse l'objet d'un contrôle afin de vérifier qu'elle n'a pas été condamnée ou mise en examen pour des infractions en lien direct ou indirect avec des activités terroristes. Par l'article 4, nous souhaitons renforcer la protection que notre pays doit aux personnes qui exercent des missions de service public face à ceux qui, par des comportements violents ou menaçants, remettent gravement en cause notre capacité à vivre sereinement ensemble. Il est urgent que nos agents publics, en première ligne face à ces dérives séparatistes, sachent que l'État sera toujours à leurs côtés et que la loi les protégera désormais plus complètement. Parce que le séparatisme use de tous les moyens pour s'étendre, ce projet de loi répond également à une menace nouvelle et pourtant déjà bien installée, qui consiste à détourner l'usage des réseaux sociaux pour les transformer en vecteur de diffusion de la haine la plus féroce et la plus décomplexée. C'est ce que nous faisons avec l'article 18 de ce projet de loi, qui crée un délit de mise en danger de la vie d'une personne par diffusion d'informations personnelles permettant son identification. L'effroyable assassinat terroriste qui a coûté la vie au professeur Samuel Paty nous l'a montré, il nous faut enrichir significativement notre arsenal législatif pour lutter efficacement contre cette haine. Pour sanctionner efficacement la volonté de nuire à autrui, le présent texte réprimera cette mise en danger, même si elle n'est pas suivie d'effet. En revanche, cette diffusion d'informations personnelles sur internet ne sera punie que si l'on démontre l'intention manifeste de l'auteur de porter gravement atteinte à la personne visée. au vu de l'expression dématérialisée et du temps de l'immédiateté, il était absolument nécessaire d'aligner le temps de la réponse judiciaire au rythme des infractions commises. C'est le sens de l'article 20, qui permettra d'ouvrir le champ de la comparution immédiate aux auteurs des propos appelant à la haine. Ce mode de poursuite permettra d'apporter la réponse rapide, nécessaire, qui fait aujourd'hui défaut à l'arsenal pénal. Il s'agit de répondre immédiatement aux discours de haine qui prospèrent aujourd'hui sur internet, notamment parmi nos jeunes, et dont les auteurs tardent trop souvent à être jugés. Cette disposition, fruit d'une large consultation organisée avec les professionnels du secteur de la presse, se fera en modifiant uniquement le code de procédure pénale. Je me félicite de ce que la rédaction proposée, et améliorée par votre commission des lois, préserve sans ambiguïté les garanties dont bénéficient les journalistes. je ne doute pas, bien sûr, de la qualité de nos débats, qui permettront sans nul doute d'enrichir ce texte. J'estime que celui-ci est absolument essentiel pour garantir l'avenir de notre pacte républicain.

l'a rappelé à l'instant le garde des sceaux, et on ne le dira jamais assez, l'école est la colonne vertébrale de la République. Comme de nombreuses institutions de la République, elle a des racines profondes, jusque dans la monarchie et l'Empire.

suffisamment large pour permettre à l'instruction en famille « normale » de continuer à être exercée. Néanmoins, nous voulons être efficaces contre les abus. Comme l'a rappelé le ministre de l'intérieur, chaque fois que nous démantelons des structures clandestines de scolarité,

voilà un peu plus d'un an que le Président de la République a placé le terme de « séparatisme » au coeur de notre débat public, une prise de conscience tardive mais nécessaire. Nous n'avions pas attendu cette parole présidentielle, toute bienvenue qu'elle soit, pour prendre la mesure du défi auquel fait face notre République. Le Sénat s'est penché, au travers de nombreux travaux, sur la question du terrorisme, sur la radicalisation, sur la place des cultes dans notre pays. Le dernier en date de ces travaux a été mené par la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre. Nous avions fait collectivement le constat de la nécessité de lutter contre la volonté d'une minorité active de soumettre à des normes prétendument religieuses la vie de nos concitoyens. Cette pression s'exerce sur les jeunes, sur les femmes, sur tous ceux que l'on veut assigner à résidence géographique ou identitaire. Pour lutter contre ce phénomène, nous avions formulé plusieurs propositions que nous sommes heureux de retrouver en nombre dans ce texte. Composé dans son immense majorité d'anciens élus locaux, le Sénat mesure la réalité de l'islam radical et de ses conséquences sur la remise en cause de l'unité nationale. Le texte que nous vous présentons est le fruit du travail de la commission des lois et de la commission de la culture du Sénat, de diagnostics de terrain et de larges concertations avec les élus, les représentants des cultes, des universitaires, des intellectuels et le monde associatif. Je souhaite rapidement vous présenter les modifications adoptées par la commission des lois sur les articles que j'ai plus particulièrement suivis. En ce qui concerne les services publics, le texte vise essentiellement à codifier de la jurisprudence et apporte peu d'innovations. Il entend inscrire dans la loi le respect des principes de neutralité et de laïcité des personnes chargées d'un service public, quelles que soient les modalités d'organisation de celui-ci. Nous débattrons du champ d'application de ce principe et des personnes auxquelles il doit s'appliquer, une question qui me semble importante. Deux catégories de personnes La première est celle des personnes qui participent de manière occasionnelle au service public. La commission des lois considère qu'elles ne sont pas toutes dans la même situation, et qu'il est en pratique impossible de leur imposer à toutes la même exigence de neutralité. nous le verrons, nous sommes favorables à aller au bout de la logique pour certaines d'entre elles, qui interviennent dans le cadre très particulier de l'école. La seconde catégorie de personnes est celle des usagers des services publics. Ici encore, nous devons être réalistes. Imposer une neutralité des usagers du service public n'a pas de sens. À l'inverse, et nous aurons ce débat, interdire, dans certains cadres délimités, le port de signes religieux ostentatoires semble S'agissant, ensuite, des mesures relatives au respect des droits des personnes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, il nous a semblé nécessaire d'être efficaces sur ces questions essentielles et sensibles, en posant des principes clairs et en ne nous contentant pas de mots. Nous avons supprimé certains articles, comme l'article 13, et en avons précisé d'autres sur les certificats de virginité ou les mariages forcés. J'en viens à la police des cultes. L'actualisation des mesures relatives à ce sujet est bienvenue, et nous la soutenons. Nous nous sommes cependant attachés à préserver la responsabilité du ministre des cultes et avons rétabli l'article 35 de la loi de 1905, en prévoyant un quantum de peine actualisé et renforcé. Par ailleurs, nous approuvons le principe d'une nouvelle mesure de fermeture administrative des lieux de culte en cas de provocation à la haine ou à la violence et avons porté sa durée à trois mois, tout en précisant les raisons pouvant conduire à cette extension. Parallèlement, nous souhaitons caractériser davantage les locaux annexes au lieu de culte qu'il sera possible de fermer s'il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de la mesure de fermeture du lieu de culte. Ces mesures pragmatiques, utiles, sont de véritables avancées dans la lutte quotidienne contre le séparatisme. J'espère que nous pourrons trouver ensemble les formulations les plus adéquates. Ce texte nous permet de donner aux services de l'État des clés et des outils nécessaires pour lutter contre le séparatisme au service de la République et de ce ciment qu'est la laïcité. Néanmoins, il ne suffira pas à construire l'immense rempart que nous avons à bâtir tous ensemble : il n'en sera que la première pierre.

vous l'avez dit, monsieur le ministre de l'intérieur, l'objectif premier de ce texte était de lutter contre le séparatisme. Mais comment y parvenir ?

Qui a combattu le plus énergiquement sa mise en oeuvre ? L'Église catholique. De 1789 à 1907, nous n'avons cessé de légiférer pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui : un État laïque qui ne reconnaît aucune religion, au sens où il les reconnaît toutes.

En 1860, le pape Pie IX spécifiait dans son les 80 propositions qualifiées d'« erreurs principales de notre temps » que Rome tiendrait désormais pour hérétiques, c'est-à-dire que celui qui les accepterait devrait abjurer sa foi. Quelles étaient ces « erreurs » ? La prépotence du pouvoir civil, la libre recherche de la vérité, les droits de la conscience, la neutralité scolaire, le droit civil, le suffrage universel, la police des cultes, la science, la liberté de la presse et de la parole, et, naturellement, l'indépendance de la morale et de la philosophie vis-à-vis du catholicisme.

Par des lois : celles de 1901, puis de 1905 et, enfin, de 1907. En 1900, Waldeck-Rousseau, qui fit voter la loi de 1901, disait Il s'agit ensuite, par la même loi, de faire face au péril qui naît du développement continu, dans une société démocratique, d'un organisme qui " tend à introduire dans l'État, sous le voile spécieux d'un institut religieux, un corps politique dont le but est de parvenir d'abord à une indépendance absolue et, successivement, à l'usurpation de toute autorité " . » La loi de 1905 se profilait déjà pour établir clairement la séparation des Églises et de l'État, c'est-à-dire du spirituel et du temporel. Je ne résiste pas à l'envie de vous préciser que c'est à Auxerre qu'Émile Combes annonça, le 4 septembre 1904, ce projet de loi. rapide avait pour but de montrer que ce que nous combattons aujourd'hui n'est pas nouveau. Il est temps de rappeler à ceux qui n'ont pas vécu cette longue histoire de séparation du spirituel et du temporel ... C'est-à-dire la ce que signifie notre laïcité, ce concept tellement français. La création de la République et la loi de 1905, cela remonte à loin dans notre monde actuel qui tend à oublier son histoire. La laïcité est notre modèle, et il faut nous en souvenir. En France, nous ne prenons pas à Dieu ce qui lui appartient, mais nous ne sommes pas prêts à lâcher ce qui appartient à César C'est pourquoi un projet de loi qui tend à inciter les associations cultuelles à respecter le régime de 1905 est utile. C'est pourquoi un projet de loi qui permet de contrôler les fonds étrangers, et donc les influences étrangères, pour nous qui nous sommes toujours battus contre l'influence du Vatican, est utile. Notre commission, monsieur le ministre, n'a donc pas bousculé votre texte ; elle l'a enrichi pour le rendre plus efficace. J'ai rappelé notre combat ancien avec les cultes, mais n'oublions pas que la loi de 1905 nous oblige. La liberté de culte est importante, et son contrôle ne peut s'exercer de façon trop tatillonne sans que nous trahissions nos propres principes. « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Aussi avons-nous fait le choix de desserrer un étau, en permettant aux préfets de s'intéresser plus directement aux associations dont le fonctionnement les interpelle lors du renouvellement de la déclaration cultuelle : cette mesure sera d'ailleurs sûrement davantage en adéquation avec les moyens dont ils disposent. En conclusion, ce texte n'est probablement pas suffisant, mais qu'il est nécessaire. J'espère donc que nos débats viendront encore l'enrichir et que les principes de notre République en sortiront réellement renforcés.

courage et lucidité : tels étaient les derniers mots du rapport de Jean-Pierre Obin en 2004 sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Dix inspecteurs généraux de l'éducation nationale pointaient déjà la « montée du phénomène religieux dans les quartiers, notamment chez les jeunes », ce qui leur valut d'être rapidement taxés d'islamophobes. Sans céder à une généralisation, les constats révélés dans des établissements scolaires constituaient les signes avant-coureurs d'une véritable lame de fond dans notre pays, dont l'école recevait déjà l'écume évolutions religieuses menant à une islamisation de certains quartiers, régression de la condition féminine, contestations pédagogiques, déscolarisations suspectes, ambiguïté voire complaisance de certaines collectivités. ans plus tard, je m'interroge sur les contours de la mission législative qui nous est confiée. Je peux reconnaître une forme de courage, au moins dans les mots, au Président de la République, qui annonçait le 2 octobre dernier aux Mureaux vouloir combattre le séparatisme islamiste. Cette idéologie qui veut imposer les lois d'une religion à celles de notre République s'illustrera de manière dramatique, quatorze jours plus tard, avec l'assassinat de Samuel Paty. Mais un combat nécessite des armes, et je doute de la lucidité des auteurs de ce projet de loi tant les moyens envisagés semblent limités au regard de l'ampleur et la profondeur du phénomène. La tumeur islamiste qui se propage au coeur de notre République a été ciblée aux Mureaux. Nous mesurons tous, je le crois, la difficulté du protocole nécessaire à son éradication, la finesse du traitement à mettre en place. Au lieu de cela, ce projet de loi prévoit d'irradier l'ensemble du corps en espérant que l'un des rayons, par un phénomène stochastique, atteindra la cible. Ainsi, la principale disposition dans le domaine de l'éducation consisterait à modifier en profondeur les modalités de l'instruction en famille cette voie d'instruction qui existe depuis trois Républiques ! Cela constitue une grossière confusion, pour ne pas dire un amalgame malhonnête, en faisant de l'instruction en famille une sorte de complice de ce séparatisme, ... Très bien ! ... alors qu'aucun élément factuel de corrélation ne m'a été présenté au cours des auditions. Outre le risque constitutionnel, le régime d'autorisation voulu par le Gouvernement instaure une suspicion généralisée à l'endroit des familles qui pratiquent l'IEF de manière régulière. Ce n'est pas acceptable, et c'est la raison pour laquelle nous avons supprimé l'article 21 en commission. Pour répondre à la problématique des enfants « hors radar » et des déscolarisations suspectes, la commission de la culture a adopté des mesures de détection différenciée afin de fermer les brèches dans lesquelles quelques-uns s'engouffrent malignement en détournant l'IEF de sa fonction première. Permettre à chaque enfant de disposer du légitime droit à l'instruction est notre priorité : c'est pourquoi nous avons créé des cellules, permis de renforcer les contrôles des inspecteurs de l'éducation nationale, ou encore interdit l'IEF aux familles dont les enfants ont fréquenté une école clandestine. Nous espérons que le Gouvernement considérera que cette démarche est à la fois plus protectrice et plus efficace. Avec l'école, le sport est l'autre entrée privilégiée du séparatisme islamiste, comme l'a montré le rapport de la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste, dont Jacqueline Eustache-Brinio était la rapporteure en 2019. Du licencié à la fédération, tous les acteurs du sport doivent se sentir concernés. C'est pourquoi la commission a souhaité renforcer la promotion des principes de la République dans le milieu sportif. L'octroi de subventions et la mise à disposition d'équipements sportifs publics seront conditionnés à l'engagement de respecter les principes de la République. Quant à l'explication de l'absence de l'enseignement supérieur dans le spectre de ce texte, j'hésite entre le manque de courage et l'absence de lucidité. L'exposé des motifs mentionne pourtant explicitement le « travail de sape » d'un « entrisme communautariste, insidieux », qui « concerne de multiples sphères [dont] les services publics ». Cet entrisme communautariste « s'invite dans le débat public en détournant le sens des mots, des choses, des valeurs et de la mesure ». Alors que de très récentes déclarations ministérielles reconnaissent l'existence d'une problématique d'entrisme islamiste à l'université, ce texte oublie un service public : celui de l'enseignement supérieur. Il faudrait nous expliquer pourquoi et comment l'université serait en dehors de notre société pour ne pas subir, comme ailleurs, les assauts du fléau islamiste. Au lieu d'être un terreau d'une extraordinaire fertilité, les campus devraient instaurer les conditions de l'éradication Nous avons donc introduit l'interdiction des prières dans les lieux inadaptés, conditionné l'octroi de locaux au respect des principes de la République, et précisé l'exercice de la liberté d'expression pour que la mission même de l'université- l'enseignement, la recherche, le débat, la confrontation d'idées

12 et 46 -, qui ont trait à son champ de compétences. Il faut noter que ces articles n'entretiennent qu'un lien assez ténu avec la lutte contre les séparatismes et le respect des principes de la République.

Ainsi, les articles 10 à 12 du projet de loi concernent l'encadrement aussi bien des avantages fiscaux attribués aux associations que de leur régime fiscal. Vous le savez, en France, les associations comme les fondations ou les fonds de dotation bénéficient d'un régime fiscal privilégié, celui du mécénat, qui permet de délivrer des reçus fiscaux aux contribuables afin de les faire bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de leurs dons.

ne faudrait donc pas que ce projet de loi, en particulier ses articles fiscaux, conduise à faire peser des contraintes trop lourdes sur ces organismes sans but lucratif, notamment sur les plus petites associations qui reposent sur le bénévolat.

qui permet d'interroger l'administration fiscale pour savoir si l'on est éligible au bénéfice des reçus fiscaux. Le recours au rescrit mécénat pourrait être d'autant plus massif que, comme la Cour des comptes l'a souligné dans un récent référé, la doctrine

L'article 11 tend à créer, quant à lui, une obligation pour les organismes sans but lucratif de déclarer chaque année à l'administration fiscale le montant global des dons et des versements dont ils ont bénéficié.

mes chers collègues, nous avons cherché en vain, dans ce projet de loi, l'équilibre du discours des Mureaux prononcé par le Président de la République le 2 octobre 2020. Plus personne ne s'en étonne, le Président qui se prétend « de droite et de gauche » marche sur la seule jambe qu'il ait jamais eue : sa jambe droite. Celle qui confond autorité avec autoritarisme, fermeté avec fermeture. Non, nous ne cédons pas à la facilité consistant à se contenter d'une société dans laquelle chaque communauté cohabiterait, même pacifiquement, côte à côte, sur un modèle anglo-saxon perpétuant des différences de droit. Nous préférons créer les conditions du rassemblement, au travers duquel peuvent s'exprimer toutes les croyances. Dans notre cité républicaine, la seule loi qui vaille est celle que les femmes et les hommes se donnent à eux-mêmes. La laïcité consiste non pas à nier la quête spirituelle chez l'être humain mais à refuser, au nom de l'unité et de la liberté, le statut politique dominateur que conférerait l'ascendant d'une religion sur la puissance publique. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est l'écart entre l'idéal républicain proclamé par le Président de la République et ce projet de loi. Non, l'exécutif ne peut pas dire, comme le fit Aristide Briand en son temps, que ce texte est un projet de loi de liberté. Du point de vue économique, les preuves d'ultralibéralisme de ce gouvernement ne sont plus à démontrer, certes, point de vue des libertés, nous ne constatons qu'un affaiblissement de nos conquêtes les plus chères. Ce projet de loi est un texte de contraintes, une addition de mesures d'ordre public : nouveaux délits pénaux, contrôle des associations, fermeture des lieux de culte. Un tiers des articles du texte instaurent des procédures de contrôle et plus d'un quart des articles définissent des peines d'emprisonnement ; même le Défenseur des droits vous en fait le reproche ! Sont pourtant concernées la loi du 9 décembre

Dès que nous sentons l'expression d'une prétendue laïcité de combat contre la religion et non contre le fanatisme, nous la combattons. Dès que la religion est manipulée par des intégristes qui ne souhaitent pas que les convictions de leurs coreligionnaires soient compatibles avec la République, nous combattons également cette dernière, il ne suffit pas d'employer la contrainte. L'exposé des motifs énonce que « la République demande une adhésion de tous les citoyens qui en composent le corps ». Je ne suis pas fin psychologue, mais croyez-vous que l'adhésion s'obtienne à coups de boutoir ? Je ne le crois pas. Il nous faut convaincre et non multiplier d'absurdes prohibitions ; l'universel doit être désiré ... Nous regrettons que ce projet de loi ne traite que les conséquences et non les causes Le phénomène dont nous parlons dépasse la question économique et sociale, mais il ne se situe pas hors du social. Il y a un séparatisme prêché par des religieux radicaux aussi un séparatisme créé par le sentiment d'abandon de certains territoires. Or le premier se nourrit du second ; c'est pourquoi un double mouvement est nécessaire : lutter contre le rejet la République, mais aussi lutter contre le rejet la République.

La contestation de la République se nourrit des signes d'hostilité et de relégation qu'adresse l'État. Il faut nous interroger sur le fait qu'une partie de nos concitoyens- une infime partie, rappelons-le -se détourne de notre modèle de société aussi facilement. Les discours hostiles à la République prospèrent le plus souvent dans des quartiers ghettoïsés, là où nous avons construit notre propre séparatisme, là où se concentrent la misère et la déréliction, dans des quartiers où la promesse républicaine n'est pas tenue, où le service public où ce recul laisse place à des organisations privées, parfois religieuses. La question n'est plus de savoir s'il faut moins d'État ou mieux d'État, un peu plus par-ci, un peu moins par-là ! Non, il faut, partout, plus, beaucoup plus d'État dans son rôle providentiel.

Nous partageons pourtant le diagnostic ; il existe un problème, que nous ne nions pas. Oui, il y a des réseaux religieux qui s'infiltrent de façon organisée dans la société, en France et dans une partie du monde, un projet politico-religieux qui conteste nos valeurs démocratiques, un projet qui vise à persuader certains de nos concitoyens de se soustraire aux lois de la République. Cela peut se manifester par la déscolarisation d'enfants, par une communautarisation de pratiques sportives ou associatives de façon générale, par des démonstrations de foi à l'intérieur d'entreprises, même chargées d'une mission de service public. Malheureusement, nous le constatons aussi, comme vous, messieurs les ministres. Nous connaissons le visage du fanatisme- ma famille politique n'a jamais fait preuve de complaisance ou de compromission lors des attentats qui ont émaillé le quinquennat précédent mais nous prétendons que le défi est encore à relever, sans angélisme, sans amalgame, sans ambiguïté face à ces forces centrifuges. certaines dispositions auraient pu emporter notre adhésion ; des sanctions plus sévères ou des mécanismes plus efficaces de contrôle des financements peuvent produire des effets bénéfiques, mais ils ne peuvent pas le faire seuls. Ce n'est pas ainsi que l'on confortera les principes de notre République. Il est facile, à l'approche d'échéances électorales importantes, de ressusciter les passions tristes. En pénétrant sur le terrain du séparatisme, le Président de la République veut apporter la preuve qu'il lutte concrètement contre ce phénomène, qu'il n'est pas naïf ; il est vrai qu'il est régulièrement accusé par la droite et par l'extrême droite d'en faire trop peu sur ce sujet. Je ne sais pas si l'extrême droite s'amollit ou si le Gouvernement s'affermit ; toujours est-il que, sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, on ne distingue plus guère la copie de l'original ... Ainsi, après ses vaines polémiques sur « l'ensauvagement » supposé de la société française, les rayons halal dans les supermarchés, sur le floutage des interventions de police et à la suite d'un essai personnel parsemé d'approximations historiques, voici le ministre de l'intérieur qui revient, avec tambour et trompette, pour expliquer aux électeurs de droite que le bulletin Macron sera plus utile que celui d'un candidat Les Républicains face à la candidate du Rassemblement national.

soit on est pour l'islamo-gauchisme. Comme il doit être reposant de considérer les choses avec cette vision binaire et simplificatrice ! Nous ne souhaitons pas participer à cette hystérisation du débat. Nous ne céderons pas à la facilité qui consiste à utiliser des abstractions pour frapper les esprits, dans une période où la politique est dominée par des objectifs de communication.

donc pas fidèle à l'« écosystème » de notre modèle. Il est paradoxal d'accorder une telle foi aux promesses d'un discours, si solennel fût-il ... Il y a beaucoup de complaisance ou de naïveté dans cet argument.

vous en déduisez l'inutilité de l'examen de ce dernier. Toutefois, vous nous permettez de retrouver ici le clivage gauche-droite. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas dupes du calendrier politique et des manipulations que celui-ci peut engendrer. Nous ne sommes pas restés béats devant ce discours, dont l'équilibre fourre-tout n'a satisfait que les admirateurs d'un « en même temps » illusoire et inaccessible. chers collègues, votre refus semble se réfugier dans l'euphémisme et il s'apparente à un véritable déni. Il est tellement difficile à expliquer qu'il masque mal vos contradictions et votre gêne. ce texte des insuffisances et des manques ; nous y voyons le moyen d'échanger, de proposer et de compléter, conformément au rôle du Sénat, sans excès, caricature ni surenchère, en veillant au respect de toutes les sensibilités de la Haute Assemblée,

qui fermons les yeux sur le refus de signer une charte d'adhésion aux valeurs de la République. Ce n'est pas nous qui flirtons avec les thèses de l'islamisme radical. Ce n'est pas nous qui voulons financer ceux qui refusent la République. Ce n'est pas nous, enfin, qui soutenons les dévoiements militants fétichisant la race Quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty et au moment de l'anniversaire de celui du colonel Arnaud Beltrame, commis le 24 mars 2018 à Carcassonne, alors que le souvenir de tous les attentats islamistes et de ses victimes nous hante- il nous poursuivra longtemps

ou- cela revient au même -vous acceptez l'idée que ce modèle n'est plus capable de se défendre lui-même. Le texte aborde une multitude de sujets, il est incomplet le Gouvernement a peut-être la main qui tremble ; mais n'êtes-vous pas concernés par les thèmes qu'il aborde : les services publics, les discriminations, l'égalité pour lutter contre différentes formes d'une inégalité homme-femme moyenâgeuse, la vie associative, les discours de haine, le libre exercice du culte, la préservation de l'ordre et de l'autorité des pouvoirs publics ? Ne voyez-vous pas que le sport, que l'on a longtemps cru protégé de tout prosélytisme religieux, est désormais le théâtre de pratiques inadmissibles et qu'il perd son rôle d'intégrateur républicain ? Ne voyez-vous pas que l'éducation subit des pratiques communautaristes qui portent gravement atteinte à ses missions et à la sécurité des enseignants ? Mes chers collègues, nous ne reconnaissons pas, dans votre refus de débattre, l'identité laïque et républicaine de certains d'entre vous, dont les partis ont dirigé la France Un mot résume votre gêne : l'émancipation. Ce mot fut longtemps, pour vous, intégré à l'idéal républicain, une émancipation souvent partagée et porteuse de progrès et de justice. Votre motion démontre que vous vous éloignez de votre propre histoire. Vous êtes à la recherche de nouvelles synthèses mobilisatrices pour votre électorat alors que vous devriez constater avec nous qu'il faut s'émanciper soi-même, à l'intérieur de la République et non être sous l'emprise de l'extérieur et d'une religion totalitaire. Ridicule ! La République ce sont des droits, ce sont des devoirs, c'est une identité, c'est la sécurité pour tous. La France doit se battre contre tous les séparatismes, notamment contre le séparatisme islamiste. L'État ne cultive aucun racisme vis-à-vis des musulmans, nous ne laisserons personne affirmer cela. Le racisme, sous toutes ses formes, doit être combattu avec fermeté. L'universalisme des Lumières nous unit pour faire progresser des valeurs communes, jamais séparées. Il faut nommer les choses. C'est l'une des grandes difficultés de l'exécutif, pris dans ses propres contradictions. Constatons ensemble que nous sommes bien en présence d'une volonté hégémonique religieuse et politique, d'un communautarisme exacerbé, dont l'endoctrinement est la matrice et le grignotage idéologique l'outil quotidien. Une religion ne peut prétendre que ses lois sont supérieures à celles de la République. Lutter contre les séparatismes n'est pas lutter contre les religions, qui doivent rester dans l'intimité de la conscience de chacun. Nous ne nous laisserons pas enfermer ou intimider et nous refuserons les débats qui veulent « cornériser » les défenseurs intransigeants de la République, les acculer dans le camp des archaïques, des anciens ou des conservateurs. Aucun tabou culpabilisateur ne s'immiscera l'intégration républicaine de nouveaux venus sur notre territoire, dans un contexte migratoire massif et non maîtrisé, pose des difficultés insurmontables, chacun le sait. Là encore, nous vous proposons la sagesse de la lucidité devant les faits. Mes chers collègues, ne vous faites pas les représentants d'une prétendue modernité, complaisante et servile ; la racialisation des problèmes sociaux et l'assignation identitaire ne représentent pas l'avenir de notre nation. La France est le fruit d'une longue histoire, sa pensée est d'une formidable richesse. Cette richesse est aujourd'hui mise à la disposition de réinterprétations, poussées à outrance, destinées à modifier nos idéaux. Les modèles venus d'ailleurs ne sont pas les nôtres ; la laïcité n'est pas négociable. Michelet l'a bien dit : « la France est une personne ».

est aujourd'hui constitué en un État dont l'unité s'est faite par l'égalité et par le mérite républicain. Notre tâche consiste à empêcher que se défassent les valeurs qui nous fondent. Mes chers collègues, la République est une volonté et une transmission. Elle est indivisible. Elle est le rempart contre l'affirmation bruyante de toutes les minorités. Elle est fondée sur ce qui rapproche les hommes et non sur ce qui les divise. Défendons la République. C'est la poursuite de la promesse démocratique qui est en jeu. À défaut, la France se condamnera à l'impuissance, au déclin, et nos concitoyens ne l'accepteront pas.

d'un seul texte, mal écrit, alternant dispositions inutiles et dispositions liberticides, quand ce n'est pas l'un et l'autre, vous foulez aux pieds les grandes lois fondatrices de la République française.

contrôle du culte. Ces lois ont été bâties grâce au compromis républicain de la fin du XIX siècle, qui avait enfin permis d'installer durablement la République dans notre pays. Elles ont été si parfaitement écrites que leur colonne vertébrale est restée inchangée depuis plus d'un siècle. Quelle arrogance, quel mépris que de vouloir en modifier ainsi la substance, sans aucun mandat du peuple ! Relisez les de Montesquieu, monsieur le ministre : « il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois. Mais le cas est rare ; et lorsqu'il arrive, il n'y faut toucher que d'une main tremblante Votre texte fait exactement l'inverse ; semblable à un marteau qui chasse une mouche, il manquera immanquablement sa cible et causera d'inutiles destructions. Il ne renforce aucun des principes républicains que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Il ne répond à aucune des problématiques qui déchirent le pacte social et nourrissent le communautarisme. la mixité sociale dans le logement ; la mixité scolaire ; tout ce qui permettrait de lutter contre la principale forme de séparatisme qui gangrène notre pays : le séparatisme social.

contribuent incontestablement à faire vivre le débat démocratique et donc à faire République. Très bien ! Depuis vingt ans, dans notre pays, la laïcité est de plus en plus instrumentalisée,

pour lequel on doit s'écouter et à propos duquel les polémiques de bas étage sont vaines, c'est bien celui-là.

Il y a des spécialistes du changement et il y a, ici, tant à droite qu'à gauche, des hommes et des femmes qui ont la fierté de défendre leurs convictions et qui savent que, lorsque l'on veut tout mélanger, on ouvre la porte aux extrémismes, car chacun a besoin de se situer, dans la République. La République a besoin non pas de confusion

si son but est de lutter contre le salafisme, contre le djihadisme radical et violent, consultez les articles du projet de loi, les uns après les autres, et citez-moi ceux qui seront efficaces à cet égard. Vous verrez que l'on accroît les contraintes en toutes choses, y compris pour les associations, sans pour autant aller dans le sens de l'objectif affirmé. Il n'y a pas de rapport entre l'objectif affirmé et les différents articles du texte. C'est pourquoi nous considérons que ce texte n'est pas bon et qu'il faut prendre les choses autrement. En conséquence, nous soutiendrons avec force la motion présentée, au nom de notre groupe, par le président Patrick Kanner.

nom des libertés. Je pense comme vous qu'ici nous devons nous respecter. C'est justement parce que chacun d'entre nous a le droit de s'exprimer et d'être libre qu'il est de notre devoir de lutter contre l'entrisme et le séparatisme.

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, en 1937, Jean Zay, ministre de l'instruction publique du Front populaire, rédigeait une circulaire, dans Je vous prie de veiller à ce que soient respectées les instructions interdisant tout port d'insignes politiques ou de propagandes confessionnelles. L'enseignement public est laïque. Aucune forme de prosélytisme ne saurait être admise dans les établissements.

Au début des années 1980 sont nés deux mouvements de jeunes antiracistes. Le premier, France Plus, avait pour mot d'ordre l'intégration républicaine et pour slogan « Nous voulons le droit à la ressemblance ». Le second, SOS Racisme, proposait le multiculturalisme. Abreuvé de subventions, surmédiatisé par tous les relais du « jacklanguisme » triomphant, il fit une entrée fracassante dans le paysage politico-journalistique. France Plus, privé de tous moyens, disparut. ans plus tard et de nombreux territoires perdus depuis par la République, la rengaine multiculturelle est partout. Le « victimisme » est devenu la base d'un discours qui aboutit, sous prétexte de tolérance, à laisser chacun à la discrétion de sa communauté, surtout des plus intégristes en son sein. Chaque jour monte un peu plus le communautarisme et, dans une certaine sous-intelligentsia universitaire, les discours délirants de l'indigénisme, de la racisation ou du décolonialisme. Les appels à la haine de soi viennent de loin. En 1961, alors que l'Afrique noire venait d'accéder à l'indépendance et que les accords d'Évian allaient être signés, Sartre écrivait : « Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé : restent un homme mort et un homme libre. Cinq ans plus tard c'est à Normale Sup qu'est apparu le spectacle effarant, au moment où le Grand Bond en avant chinois faisait 50 millions de victimes, de centaines d'étudiants brandissant frénétiquement le ridicule, pendant qu'à Pékin des millions de Chinois étaient forcés, eux, de le faire sous peine de mort. Un sot savant est plus sot qu'un sot ignorant » disait Molière. Aujourd'hui, c'est des facultés de sciences humaines que de pâles copieurs de campus américains devenus fous nous proposent la version XXI siècle de l'extrémisme déjanté. Après l'apologie du stalinisme, du trotskisme, du maoïsme, du tiers-mondisme, de l'altermondialisme, du collaptionisme, voici venir l'éternel retour du même sous la forme de l'indigénisme et de l'islamo-gauchisme. Frédérique Vidal a eu le mérite de nommer l'éléphant que personne ne voulait voir dans les locaux universitaires. Mais quelle idée d'en proposer l'étude au président du CNRS,

Dans une société non métissée, le social et le genre dominent, mais dans l'espace interracial, le social s'efface derrière le racial. » Il s'agit bien du président du CNRS ... C'est un peu comme si l'on confiait au cow-boy Marlboro une enquête sur les méfaits du tabac. Il a répondu à la ministre que l'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique. C'est un peu bizarre pour un concept forgé en 2004 par Pierre-André Taguieff, directeur de recherche au CNRS. pour le président du CNRS d'aujourd'hui, le « racisme d'État », le « privilège blanc », la « culture du viol » et la « fluidité identitaire » semblent être le des concepts scientifiques. On attend impatiemment les résultats de l'enquête Est-ce « islamo » ou est-ce « gauchisme » que l'éminent scientifique a du mal à comprendre ? C'est pourtant simple : islamo est la contraction d'islamisme ; gauchisme, c'est gauchisme. Islamo-gauchisme, c'est quand le gauchisme fricote avec l'islamisme.,

Au sujet de l'UNEF, le professeur Mélenchon, souvent dans l'erreur mais jamais dans le doute, a écrit mardi dernier sur son blog : « Défendre l'UNEF, c'est lutter contre l'obscurantisme. » Sans commentaire. Cette manifestation maigrelette fut pourtant un événement considérable, parce qu'elle a consacré la fracture de deux gauches. D'un côté, la gauche restée fidèle à ses idéaux laïques et républicains, inflexible sur la mise à distance des assignations identitaires de l'autre, la gauche des idiots utiles de l'islamisme qui espèrent enrôler les musulmans dans leur combat intersectionnel, dont, pourtant, la quasi-totalité des musulmans ne veut pas. On pourrait penser que je me réjouis de cette fracture, qui risque d'assurer à la gauche de longues vacances. Mais je ne m'en réjouis pas, car, avec la pression croissante de l'islamisme et du communautarisme, l'unité nationale autour de nos principes est cruciale. Et dans cette guerre des deux roses, j'ai peur que la dynamique et le battage médiatique ne soient pas, hélas, du côté de ceux qui défendent la laïcité- semblent, avec cette question préalable, avoir un petit coup de mou cette après-midi. Il est plus que temps de s'attaquer à la montée des séparatismes, des fondamentalismes et des projets antirépublicains. C'est ce que vous nous proposez aujourd'hui, messieurs les ministres et il n'y a pas de raison de ne pas vous suivre. pas vous suivre. Mais, vous le savez, il y faudra beaucoup plus qu'une loi. Il y faudra une volonté. C'est sur elle que vous-mêmes, votre gouvernement et nous-mêmes parlementaires serons jugés.

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, penchons-nous sur l'exposé des motifs de ce texte. Qu'y lisons-nous ? « Un entrisme communautariste, insidieux mais puissant, gangrène lentement les fondements de notre société dans certains territoires. Cet entrisme est pour l'essentiel d'inspiration islamiste. Il y a peu, Mme Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur déclarait, elle, que l'islamo-gauchisme « gangrénait » la société. La récurrence de ce terme médical n'est pas anodine. Elle en dit long sur la perception que certains ont, en France, de l'islam. Celui-ci infecterait, pourrirait, rongerait notre pays. Au lieu de proposer des solutions pour contrer l'islamisme radical en agissant efficacement dans les territoires touchés et en mettant à la disposition de cette action tous les moyens publics nécessaires, ce texte ne suggère que de couper des membres gangrénés. pas, bien sûr, à faire cesser, dans l'esprit de trop de nos concitoyens, la confusion entre islamisme radical et islam. Élaboré après l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, ce texte, dont plus d'un tiers des articles vise à renforcer les dispositifs de contrôle et près d'un quart définit des peines d'emprisonnement, facilitera-t-il la lutte contre le mal qu'il dénonce ? Je crains que non et je suis la première à le regretter. Il tend surtout à renforcer le contrôle social, à restreindre les libertés et à réprimer tout ce qui ne se soumet pas à l'ordre social que le pouvoir appelle de ses voeux en cette veille d'élection présidentielle, espérant ainsi récolter des voix à la droite et à l'extrême droite. Ses répercussions seront, de surcroît, importantes sur la vie des autres cultes. L'archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France, m'écrivait dès janvier : « Pour le dire synthétiquement, la loi de 1905 est une loi de liberté. Elle risque, avec ce projet de loi, d'être transformée en une loi de contrôle, de police et de répression. » Il ajoutait Pour acquérir des moyens nouveaux d'empêcher les islamistes radicaux de mener à bien leur projet, l'État multiplie les contrôles et organise une nouvelle mise sous tutelle des cultes. Je le rappelle, c'est un archevêque qui parle, pas la Défenseure des droits. Le Conseil d'État juge lui-même que « le projet de loi alourdit les contraintes pesant sur les associations cultuelles et modifie l'équilibre opéré en 1905 par le législateur ». Ce texte consacre en fait, pour reprendre les mots de François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France, « la dérive progressive et inquiétante de la compréhension de la laïcité comme la grande idée libérale de 1905 vers une neutralisation religieuse de notre société ». Les libertés associatives sont globalement menacées par ce texte. Les associations, même non religieuses, s'en inquiètent. Elles voient l'octroi de subventions conditionné à la signature d'un contrat d'engagement républicain aux contours flous et à l'engagement de s'abstenir de toute action préjudiciable à l'ordre public. Les associations écologistes pourraient bien, à terme, en pâtir à leur tour. Car il s'agit bien d'un texte de suspicion généralisée. Ses cibles sont aujourd'hui musulmanes. Elles pourraient bien se diversifier à l'avenir. La laïcité, socle de notre cohésion nationale, n'est plus ici qu'un prétexte pour bâtir une République autoritaire et intrusive. Dans un pays sous état d'urgence sanitaire depuis plus d'un an, M. Darmanin transforme notre pacte républicain en une chape répressive. L'article 18 relatif au délit de mise en danger de la vie d'autrui par la diffusion ou la transmission d'informations sur internet, de l'ancien article 24 de la proposition de loi, dont le nouveau titre est « Pour un nouveau pacte de sécurité respectueux des libertés », l'atteste bien. Ce projet de loi s'intitule lui-même « Respect des principes de la République ». Respect », « respectueux », voilà des mots qui disent le contraire de ce que ces textes sont vraiment : liberticides. Il est à regretter que les principes étriqués de la République macronienne prennent le pas sur l'esprit de de nos lois, loi de 1905 comprise. Le combat contre le fanatisme de certains groupes islamistes et contre le terrorisme est également notre combat, mais pas en obtempérant obtempérant à ce texte. Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ne pourra que voter contre ce texte. La parole

nous ne pouvons ouvrir ce débat sans nous accorder sur un diagnostic partagé. Le constat qui, je crois, peut nous rassembler, au-delà de la terminologie qu'on entend lui rattacher, est celui d'une force de fragmentation exercée par des lois particulières sur la norme commune. Il ne s'agit pas ici de défendre l'idée que les lois particulières, spirituelles notamment, porteraient en leur nature la faction, la séparation ou la sécession. Il faut le redire, ce projet de loi n'est pas animé par une défiance envers le fait religieux ni, bien sûr, à l'égard de la démarche associative. Non, il relève d'une stricte ambition de répondre aux pressions de morcellement de la société, aux volontés d'une fraction extrémiste de la population de quitter la République et aux différentes assignations et menaces mortifères auxquelles ces désagrégations conduisent. Ce constat d'une dynamique de fragmentation, une fois posé, doit nécessairement être dépassé pour trouver les modalités de réponse que le législateur peut lui apporter. La tâche n'est pas aisée : non seulement la réponse ne saurait être simple et univoque, mais elle n'est pas non plus réductible à un véhicule législatif. Il apparaît, en tout cas, que la voie empruntée par le texte, dans la continuité des discours de Mulhouse et des Mureaux du Président de la République, ne remet pas en cause les libertés dont il est question. Je pense à la liberté d'association et au principe de laïcité, clé de voûte, en creux, de la loi du 9 décembre 1905 et dont découlent la liberté de conscience et le libre exercice des cultes ainsi que la neutralité de l'État. Je pense également à des principes matriciels, tels que l'universalisme et la conception élective de la Nation, ce « plébiscite de tous les jours », pour reprendre les mots éclairants d'Ernest Renan. L'inscription dans la continuité des législateurs du début du XX siècle est soulignée par le Conseil d'État. Nous retrouvons cette continuité dans plusieurs des dispositions du projet de loi, telles que la possibilité pour les associations cultuelles de posséder et d'administrer des immeubles de rapport acquis à titre gratuit ou encore le maintien de la liberté, pour les cultes, de choisir les modalités de recrutement de leurs officiants et de s'organiser sous trois régimes différents. Cela, conformément à la loi de 1907, et en procédant plutôt par un mécanisme d'incitation à rejoindre le régime de l'association cultuelle. D'autres dispositions utiles du projet de loi ont été conservées en commission. Je citerai : les mesures de transparence des financements étrangers les articles relatifs au service public, avec notamment le nouveau délit de séparatisme ; le contrat d'engagement républicain ; le renforcement de la lutte contre la haine en ligne, en cohérence avec la dynamique européenne ; ou encore la garantie de la dignité de la personne humaine au travers de l'égalité femmes-hommes. Je n'oublie pas, bien sûr, la partie relative à l'application des dispositions en outre-mer : elle ne remet pas en question- c'est heureux -les équilibres de ces territoires, notamment en Guyane et à Mayotte. Le texte va évoluer sous l'effet de nos débats et de nos initiatives. Certains des amendements en commission sont d'ailleurs venus utilement consolider le texte ou prévoir des assouplissements, et j'en remercie nos corapporteures. Je pense à l'explicitation du champ d'application des nouvelles obligations des associations mixtes. Plusieurs débats vont animer notre hémicycle- ils ont d'ailleurs déjà commencé -, notamment la question du champ d'application de l'obligation de neutralité et le sujet du port des signes religieux. Sans préjuger de leur issue, j'aimerais toutefois rappeler que, lors de l'examen en commission, plusieurs propositions allant dans ce sens ont été rejetées sur le fondement d'une question méthodologique simple, mais indispensable les dispositions sur lesquelles nous nous prononçons permettent-elles d'atteindre le but, que nous partageons, de renforcer le respect, par tous, des principes de notre République ? À la lumière de cette question, que nous nous sommes posée collectivement en commission, l'absence de certaines dispositions dans le texte procède, je crois,

mes chers collègues, que Charb entamait son discours de remise du prix 2012 de la laïcité, décerné à notre ancienne collègue Françoise Laborde. Il poursuivait ainsi : « Et j'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïques qui se taisent. » tonnerre d'applaudissements, à l'époque, avant que le silence ne reprenne sa place et que la dénégation ou le manque de courage ne fassent leurs ravages. Car, malgré le choc des attentats de 2015 et la disparition de tant d'innocents, dont le dessinateur, petits arrangements et contournements ont repris de plus belle. Nous avons laissé s'exprimer, certes parfois en nous agitant mais jamais assez fort, ceux qui disent qu'« après tout ils l'ont bien cherché avec leurs caricatures laissé dire ceux qui affirment que l'engagement de nos troupes militaires à l'étranger est une provocation permanente. Nous avons laissé dénoncer ceux qui prétendent que nos lois sont finalement liberticides et islamophobes. Nous avons permis à ces bruits de fond de parasiter depuis des années notre société et à ces attaques insidieuses et pernicieuses de saper notre modèle laïque. La sentence tombe tel un couperet : comme moi, vous avez découvert, atterrés, les conclusions de l'enquête IFOP pour la Ligue sont implacables : nos jeunes sont majoritairement favorables à l'expression de la religiosité dans l'espace public et hostiles à la liberté de la critique des religions. Combien d'entre eux sont persuadés que le blasphème est un crime en France ? Comment en sommes-nous arrivés là ? En consacrant la séparation des Églises et de l'État, la loi du 9 décembre 1905 a fondé notre ordre démocratique, forgé notre pacte républicain et étayé notre devise à l'équilibre si fragile. Pourtant, la défendre aujourd'hui c'est mettre sa vie en danger. Nous l'avons subi avec de trop nombreux crimes jusqu'à l'assassinat récent de Samuel Paty, professeur des collèges. Depuis ce drame, le Président de la République a enfin amorcé la sortie de ce long déni collectif politique et intellectuel. Mais combien d'années se sont écoulées avant de nommer l'ennemi et l'identifier correctement ? On nous a parlé de terrorisme, de communautarisme, de radicalisme et maintenant de séparatisme. Or le définir, c'est le connaître, le suivre et lutter contre le coeur de son action.

Aux côtés de la rapporteure Jacqueline Eustache-Brinio, que je salue, j'ai eu l'honneur de présider ces travaux visant à susciter une prise de conscience rapide et clairvoyante. Notre objectif partagé était de démontrer l'ampleur du phénomène de radicalisation au-delà de ses seules manifestations violentes. Nous avons mené plus de soixante heures d'auditions pour identifier consciencieusement les dérives observées sur notre territoire, sans préjugé ni tabou. Face à l'urgence, nous avons éclairé les secteurs devant faire l'objet d'une vigilance particulière, comme l'enseignement, le monde associatif ou encore sportif, dans lesquels la pression séparatiste est forte. Nous retrouvons ces secteurs dans ce texte, même si force est de constater que notre école publique et nos établissements d'enseignement supérieur ont été ici quelque peu mis de côté. Je salue donc les amendements portés par la commission de la culture et de l'éducation pour corriger cet écueil. regrettable, monsieur le ministre de l'éducation, que vous ayez déporté le débat sur l'instruction en famille (IEF). En stigmatisant l'IEF, vous avez choqué des milliers de parents qui ont fait ce choix alors qu'ils ne remettent pas en cause notre pacte républicain. Les priver de cette liberté, c'est faire le jeu des islamistes et les laisser remporter une victoire de plus. Permettez-moi de vous rappeler que, dès février 2019, j'ai déposé- vous le savez -une proposition de loi, qui fut portée par amendements lors de la loi pour une école de la confiance aux fins de combattre les dérives que vous dénoncez depuis peu. Ces amendements visaient à améliorer à améliorer l'identification l'identifiant national élève (INE) généralisé, le contrôle et le suivi de ces enfants, sans entraver la liberté de choix d'instruction des parents. Vous les aviez balayés et, aujourd'hui, vous vous en inspirez. Nous avons perdu deux ans. difficile de ne pas souligner l'absence de mesures adressées au monde économique, qui fait pourtant face aux mêmes problématiques. Pour preuve, le nombre de saisines de la Défenseure des droits témoigne de la dégradation de l'ambiance dans nos entreprises. Je regrette aussi que nos élus locaux n'aient pas bénéficié d'un arsenal de mesures dédiées pour les accompagner dans la gestion des relations avec les représentants religieux et mettre fin à toute forme d'accommodement local. Des 44 propositions contenues dans notre rapport sénatorial publié le 7 juillet dernier, de très nombreux dispositifs ont été transposés dans votre projet de loi.

que me réjouir que nos travaux aient pu s'incarner dans ce texte, faute d'avoir été salués. Je pense à des mesures comme le renforcement de la police des cultes, l'alignement des statuts légaux et fiscaux des lois de 1901 et de 1905, le prérequis d'une charte pour le versement de subventions, le régime de déclaration des apports de ressources étrangères, etc. Je remercie également la commission des lois d'avoir adopté des dispositifs complémentaires défendus par la commission d'enquête : la dissolution administrative d'associations placée sous le contrôle du juge administratif l'intégration du sexe ou de l'orientation sexuelle dans le champ des motifs de dissolution, ce qui devrait permettre de viser des structures soutenant la lapidation des femmes ou la mise à mort de personnes homosexuelles le renforcement des sanctions en cas d'atteinte à la liberté d'exercer un culte ; ou le dispositif visant à mieux protéger les conjoints et les mineurs. Messieurs les ministres, défenseur des acquis de la loi de 1905, le RDSE présentera, tout au long des débats, de nombreux amendements visant à préserver cet héritage et faire de la laïcité notre meilleure arme contre le radicalisme religieux pour que notre pacte commun en sorte réaffirmé, que notre socle de valeurs s'en trouve consolidé et qu'enfin seules les lois de la République prévalent ! La parole

de loi dont nous entamons l'examen aujourd'hui répond-il aux attentes de nos compatriotes ? Ce texte, qui a pour objectif affiché de lutter contre l'influence de l'islamisme politique dans notre société, est-il d'une telle urgence qu'il faille en discuter en procédure accélérée plutôt que de traiter les besoins qu'exprime notre peuple face à la crise sanitaire ? ? Oui, bien sûr, l'évolution du monde et la dégradation profonde de notre tissu social nourrissent le développement d'un fondamentalisme. Celui-ci s'appuie, en la détournant, sur la religion musulmane pour imposer, dans des pays, des régions du globe, mais aussi dans des quartiers, une conception politique, que je qualifierais de « fascisante », de la société. Je vous le dis d'emblée, ce n'est pas par l'empilement de règles plus répressives les unes que les autres que vous répondrez à la déshérence d'une population qui ne croit plus forcément à la République, car celle-ci l'a délaissée. L'urgence est ailleurs aujourd'hui. L'urgence est d'aider l'hôpital. L'urgence est de restaurer notre capacité à produire des vaccins. L'urgence est d'agir pour le climat. L'urgence est de venir en aide aux 10 millions de pauvres dans notre pays Ce qui doit être éradiqué dans l'immédiat, c'est le malaise étudiant, la détresse sociale, la faim, et certainement pas le fantasme d'un islamo-gauchisme, concept que le Gouvernement, Mme Vidal en tête, et d'autres ici encore aujourd'hui livrent en pâture à l'extrême droite. L'urgence, ce sont les plans sociaux, toujours plus nombreux. Or, pour le Gouvernement, l'urgence des urgences est de légiférer sur le séparatisme islamiste. L'évolution d'Emmanuel Macron est patente

La notion de séparatisme ne figure plus dans l'intitulé du projet de loi, et pour cause : le grand texte relatif au séparatisme en matière de religion est celui de 1905, qui assura la séparation de l'Église et de l'État et qui acta l'entrée de notre pays dans une République laïque, après une longue histoire. Le mot « séparatisme » se perd finalement dans les contradictions fondamentales de votre action. De surcroît, vous ne pouvez pas défendre ce concept alors que le séparatisme fondamental de notre société est aujourd'hui celui des riches avec les pauvres. Notre pays subit de plein fouet un séparatisme multiple : séparatisme scolaire, séparatisme universitaire- 30 % des enfants de classes défavorisées intégraient l'ENA, l'ENS ou HEC en 1950, aujourd'hui -, séparatisme territorial, renforcé par la mise à mal de l'unicité du service public dans notre pays. Avec votre texte, le discours prononcé par Emmanuel Macron aux Mureaux en octobre dernier paraît bien loin. Le Président de la République, comme à son habitude, avait prôné le « en même temps » : il faut réprimer le séparatisme islamique, mais il faut aussi restaurer la République sur tout le territoire. Je le cite Nous avons nous-mêmes construit notre propre séparatisme. C'est celui de nos quartiers, c'est la ghettoïsation de notre République [ ...] Nous avons construit une concentration de la misère [ ...] Nous avons créé ainsi des quartiers où la promesse de la République n'a plus été tenue. » M. Macron a jeté aux orties l'habillage social de son propos pour ne conserver que l'objectif répressif et coercitif. Nous nous trouvons donc face à un texte présenté comme l'héritage des auteurs de la loi de 1905, alors que celle-ci était fondamentalement une loi de liberté. Dans son article 1, elle garantit la liberté de conscience et la liberté des cultes, et, dans son article 2, elle affirme La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. » C'est la séparation de l'Église et de l'État, à l'opposé d'une démarche concordataire qui subsiste encore en Alsace-Moselle, avec les récentes conséquences que nous connaissons, et dans quelques autres départements et territoires.

votre texte déborde la question religieuse. Il instaure un contrat d'engagement républicain. Là aussi, qui le définit ? Qui le valide ? Vous placez l'ensemble des associations sous tutelle. Vous rétablissez le lien entre l'État et les religions, alors que, vous le savez bien, l'ensemble des associations cultuelles critiquent cette évolution. Vous remettez en cause la liberté d'association, en plaçant au coeur d'un contrat d'engagement républicain la question du respect de l'ordre public. Regardons le contrôle du financement des associations culturelles. M. Patrick Weil affirmait fort justement : « La loi prévoit déjà depuis 1905, pour les associations culturelles, le contrôle de l'administration fiscale et de l'inspection générale des finances. Les contrôles ont-ils été faits quand ils auraient dû l'être ? C'est la maladie française. On fait des lois pour camoufler l'absence d'action dans le cadre des lois précédentes. »

Je ne supporte pas la stigmatisation dont sont victimes les millions de musulmans ou celles et ceux que l'on considère comme tels, qui habitent dans notre pays et dont la très grande majorité sont nos compatriotes. Je ne supporte pas que, pour une minorité agissante, qu'il faut combattre- les communistes n'ont jamais failli à ce combat et l'ont trop souvent payé de leur vie dans des pays où les guerres civiles firent rage -, une part significative de notre peuple soit montrée du doigt. Ma colère, monsieur le ministre de l'intérieur, est d'autant plus vive que ces femmes, premières victimes de tous les obscurantismes, et ces hommes sont souvent confrontés à de grandes difficultés sociales. Je ne peux accepter ce que vous avez écrit dans votre livre à propos de ceux qui s'inquiéteraient d'une « xénophobie d'État », stigmatisant ceux « qui mêlent leurs voix et leurs protestations aux cris et aux actes de ceux qui attaquent la France » et qui seraient- je vous cite encore

le 2 octobre dernier, le Président de la République a tenu un discours important sur la lutte contre les séparatismes. Le 16 octobre, soit quatorze jours plus tard, Samuel Paty était assassiné par un terroriste islamiste dans les rues près de son collège. Ces circonstances nous obligent, et ce n'est pas, monsieur Grosperrin, nous référer béatement à un discours du Président de la République que de considérer que, le jour où le chef de l'État s'exprime sur un sujet aussi grave, il est important de l'entendre, de le lire et de nous demander quelles conséquences nous pouvons en tirer. Dès lors, je vous le dis, je trouve inacceptable

Pour la gauche, la République doit être la République « jusqu'au bout », pour reprendre la formule de Jaurès, avec l'ordre républicain d'un côté et la promesse républicaine de l'autre. est fondamentalement attaché au respect des principes de la République et à leur protection. Nous saluons les femmes et les hommes qui la servent : fonctionnaires, militaires, enseignants, personnels soignants ... Nous saluons tous ceux qui ont choisi de servir l'intérêt général. Nous sommes attachés à la laïcité. Oui, nous sommes fidèles à l'héritage de Jaurès, de Briand ou de Ferdinand Buisson, à cette liberté de croire ou de ne pas croire. Et nous sommes attachés à la dignité humaine, contre toutes les pratiques indignes, en particulier contre les femmes.

la République était à la fois un ordre et une promesse, mais il a évoqué un « devoir d'espoir » et le besoin de « faire aimer la République » pour que chacun « puisse trouver sa place. » Or cette seconde partie du discours du Président de la République a disparu : pas un mot sur la mixité sociale, sur la discrimination en matière d'emploi ou de logement, sur l'accès aux services publics ou encore sur l'égalité des chances. Or la République est une promesse : la promesse d'être intégré, de participer. C'est la promesse républicaine d'égalité et d'émancipation. Les élus locaux que nous Nous savons que, si nous n'abordons pas ces sujets, le texte est totalement déséquilibré. Or, dans ce texte, notre République est réduite à des règles, à des interdictions, à des motifs d'ordre public. Nous n'y retrouvons pas le pendant que constituent les droits, l'égalité, la solidarité et les principes de la République. De toute

créera une concurrence juridique qui rendra très complexe la poursuite des infractions. Je pense que le Gouvernement devrait y veiller. Ce texte est aussi un texte de défiance, envers les croyants, les membres d'associations, l'école et, au final, tous les citoyens. Comme si chacun devenait suspect et allait se radicaliser ... Sur quelques points, nous partageons les dispositions de ce projet de loi. Par exemple, nous souscrivons aux mesures permettant une meilleure protection des agents du service public ou à celles qui visent à améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes. L'interdiction des certificats de virginité, la lutte contre les mariages forcés ou la polygamie sont des combats que nous partageons évidemment et sur lesquels mes collègues Jacques-Bernard Magner et Jean-Pierre Sueur reviendront tout à l'heure. Mais, comme vous l'aurez compris, nous ne nous satisfaisons pas de l'ensemble de ce projet. En quoi pourra-t-il enrayer la fuite hors de la société de certains, le repli sur soi, l'entre-soi ? Pourrons-nous mieux vivre ensemble quand il Les Français seront-ils mieux protégés ? Allons-nous restaurer cette République, qui permet et promet tant ? Ces sujets auraient dû être abordés d'une main tremblante, comme le disait Montesquieu, car on ne peut sans conséquence modifier des textes fondateurs comme la loi de 1905 ni légiférer sur des questions aussi fondamentales. Il est incontestable que, lors de la rédaction de ce texte, la main du Gouvernement n'a pas tremblé suffisamment. Aujourd'hui, au Sénat, nous devons appréhender ce texte comme il aurait dû être rédigé un texte d'ordre, sans doute, mais aussi comme un texte de promesses, ce qu'il n'est pas. Vous l'avez compris, nous n'approuvons pas ce texte.

M. Stéphane Ravier. Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, « dans vingt ans, c'est sûr, la France sera une République islamique Tel était le voeu exprimé en 1986 dans le par un certain Hussein Moussaoui, l'un des chefs du Hezbollah libanais. Si, trente-cinq ans plus tard, ce projet n'est pas achevé, force est de constater qu'il est en cours de réalisation, car ce ne sont pas moins de 150 quartiers en France qui sont aujourd'hui tenus par les islamistes. Et ces quartiers ne se situent pas seulement dans le secteur nord de Marseille, dans la banlieue lyonnaise ou parisienne. On en trouve aussi à Annemasse, à Lunel, à Oyonnax, à Nogent-le-Rotrou ou encore à Maubeuge, où le clair de lune a été remplacé par le croissant de lune islamique. Et ce n'est plus du tout la même chanson ... Pendant ce temps, votre gouvernement, messieurs les ministres, n'a toujours pas le courage de nommer le mal. Cette frilosité vous conduit à des contorsions sémantiques et législatives, qui ne sont pas sans conséquences sur les libertés publiques en général et sur les libertés des autres religions en particulier. Faute de nommer l'ennemi, votre texte est liberticide pour ceux qui respectent la loi et largement insuffisant pour ceux qui la piétinent.

Et, puisque les choses doivent être dites, ce ne sont pas tant les valeurs de la République que les islamistes veulent abattre que la France : la France des terroirs et des clochers, la France enracinée, la France française Aujourd'hui, en France, 57 % des jeunes musulmans préfèrent l'application de la charia- la loi islamique -aux lois de la République. Plus d'un jeune musulman de France sur deux ne se reconnaît donc pas dans le modèle qui l'a vu naître. Ils n'ont que faire de votre vivre-ensemble ! Ils ne sont même plus dans la séparation : ils sont dans une volonté de conquête, exigeant que nous vivions comme eux. Les métastases islamistes se sont répandues dans tout le corps national. Elles ont contaminé nos écoles, nos universités, nos médias, la culture, le sport et, même, et, même, nos hémicycles. Et la majorité écrasante des terroristes sont des étrangers ou des produits issus de l'immigration. De fait, je n'aurai de cesse de le répéter, l'islamisme n'est pas une cause : c'est une conséquence de l'immigration massive. Après avoir nommé le mal et identifié ses origines, sachons nous attaquer à ses soutiens de l'intérieur. Le poisson, y compris politique, pourrit toujours par la tête. Les islamistes savent pouvoir compter tant sur l'islamo-gauchisme que sur l'islamo-droitisme, le premier par idéologie antifrançaise et le second par électoralisme, lequel conduit nombre d'élus locaux à collaborer avec l'ennemi. obtenir 51 % des voix, comme d'autres voulaient trente deniers, on fait subir à la France, aux Français et à notre civilisation européenne un véritable calvaire. Le texte du Gouvernement est une occasion ratée de vacciner notre pays contre la pandémie islamiste. Je vous engage dès lors, mes chers collègues, à soutenir les initiatives visant à lui donner toute la force et la détermination dont il a besoin. L'avenir n'est jamais irrévocable : il sera ce que nous aurons décidé. Dans tous les cas, soyez assurés qu'il vous jugera

Il pose, en filigrane, une question centrale : face à la transformation de nos sociétés, où nous perdons de vue ce qui nous est commun au profit des droits individuels, comment concilier la liberté du citoyen et celle de l'individu ? ? Un cadre juridique existe. Il est parfois paradoxal. L'article 1 de notre Constitution énonce que la République laïque respecte toutes les croyances. La laïcité est le fruit d'un long débat. Elle résulte d'un compromis. La loi de 1905, vécue douloureusement, s'inscrit dans un contexte de lois antérieures antireligieuses. Elle a été voulue comme une loi d'équilibre, tenant compte de la réalité de la société française à cette époque. Un écart, parfois considérable, existe entre le principe recherché et la réalité. La laïcité, telle qu'elle s'est construite, est une réalité historique, définie en fonction des situations et des problèmes rencontrés. Il en est ainsi aujourd'hui avec une religion qui, en France métropolitaine, n'existait pas au début du siècle dernier. Les acteurs du débat d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes, leurs références non plus. De même, la notion de laïcité peut ne pas recouvrir la même signification selon les générations. La méthode qui a présidé au début du siècle est celle de l'apaisement, pour « la liberté dans la diversité », comme le plaidait Clemenceau, et la République « cité des consciences autonomes », selon le philosophe Charles Votre projet de loi, monsieur le ministre, s'efforce à l'équilibre. Il le revendique. L'islamisme politique et le salafisme se nourrissent de l'inorganisation de l'islam en France. C'est une part importante du sujet. Mais la loi ne peut contraindre une religion à s'organiser. D'un côté, il nous faut lutter contre la propagation du séparatisme, contre la haine en ligne, pour la protection des services publics, pour l'incitation des cultes à intégrer le statut de la loi de 1905, et connaître leurs financements afin de s'assurer de l'absence de toute ingérence étrangère. faut pas attenter à la liberté de culte, à la liberté d'expression, à la liberté de religion, à la liberté d'association, avec pour seuls outils la loi égale pour tous, l'ordre public, les règles minimales de vie en société, l'intérêt public local, l'intérêt vital de la Nation. La commission des lois a, je le crois, permis d'aller plus loin dans l'équilibre, jusqu'à ce matin. J'espère que ce mouvement sera constant. Je rejoins de nouveau Clemenceau, qui déclarait : « S'il devait y avoir un conflit entre la République et la liberté, c'est la République qui aurait tort. Concernant la neutralité des services publics, notre commission s'est montrée cohérente en étendant aux salariés participant à une mission de service public les mêmes obligations que les agents publics et a refusé leur extension aux élus au-delà de leurs fonctions d'agent de l'État. Elle a amélioré le contrat d'engagement républicain, en transférant au préfet l'obligation d'informer les organismes qui concourent au financement d'une association s'étant vu retirer une subvention, alors que les députés avaient confié cette obligation aux élus locaux.

Concernant le respect des droits des personnes et l'égalité entre les femmes et les hommes, nous soutenons les articles qui interdisent la polygamie et qui prohibent et pénalisent la réalisation par des professionnels de la santé de certificats de virginité. De même, nous sommes favorables au dispositif de lutte contre l'excision. La commission a fait oeuvre utile concernant les mariages forcés ou viciés, en prévoyant que l'officier d'état civil puisse consulter une base de données nationale recensant l'ensemble des décisions d'opposition et de sursis à mariage.

La commission des lois a amélioré l'équilibre entre liberté de culte et nécessaire contrôle, notamment des financements, sans pénaliser les associations qui sont respectueuses des lois de la République. Nous pouvons encore apaiser et améliorer l'équilibre et rendre plus attractif le cadre de la loi de 1905. Par exemple, pour rendre davantage autonomes les associations cultuelles dépourvues de financements étrangers, la commission a supprimé le plafond de 33 % que devaient représenter les ressources tirées d'un immeuble acquis à titre gratuit. Nous sommes nombreux à vouloir que les associations puissent également vivre de ressources issues d'immeubles acquis à titre onéreux. Comme l'a souligné Philippe Bas, il est incompréhensible aujourd'hui en l'absence de toute capacité immobilière, les associations cultuelles puissent placer leurs trésoreries dans un portefeuille d'actions, mais qu'elles n'aient pas la possibilité d'acheter un immeuble. De même, toujours dans un souci d'autonomie financière des associations cultuelles, nous avons, avec mes collègues, déposé un amendement visant à augmenter le plafond des dons en liquide pour l'aligner sur celui qu'a prévu le décret de 2015 concernant le paiement en espèces entre particuliers et professionnels. Enfin, s'agissant des dispositions relatives à la police des cultes, si la commission a approuvé le nouveau dispositif de fermeture administrative des lieux de culte en cas de provocation à la haine ou à la violence, elle a limité à trois mois la durée de cette fermeture. Ce dispositif est apparu disproportionné à certains, car il n'est pas assorti de garanties telles que le contrôle par le Parlement sur la base de rapports réguliers présentés au Sénat et à l'Assemblée nationale. Dès lors, il paraît attentatoire aux libertés publiques. Nous souhaitons le limiter dans le temps. C'est l'objet de l'amendement n° 584 rectifié. Pour conclure, je citerai Locke, dans sa, en 1686, écrivait : « Il est d'une nécessité absolue de distinguer ici, avec toute l'exactitude possible, ce qui regarde le gouvernement civil, de ce qui appartient à la religion, et de marquer les justes bornes qui séparent les droits de l'un et ceux de l'autre. Sans cela, il n'y aura jamais de fin aux disputes qui s'élèveront entre ceux qui s'intéressent, ou qui prétendent s'intéresser, d'un côté au salut des âmes, et de l'autre au bien de l'État. » Apaisons, équilibrons encore Mesdames les rapporteures, je salue votre travail et celui qu'il vous faudra encore réaliser dans les débats à venir. Apaisons, équilibrons encore, sans empêcher évidemment que la cible soit bien atteinte. Très bien ! La parole est à M.

est la suivante : le courage est-il au coeur du texte ? Nous le savons, la situation est gravissime. Tous les sondages, toutes les études nous le démontrent. Aurons-nous le courage qu'impose la difficulté de la situation ? J'aurais, monsieur le ministre, aimé répondre « oui

vous n'allez pas au bout des choses quand vous vous arrêtez à mi-chemin sur la neutralité et sur la laïcité. Vous n'osez pas parler du voile. Dans notre histoire récente, des gouvernements ont fait un autre choix,

cet ennemi a une histoire, une mémoire, un récit. Il voudrait ramener nos compatriotes français musulmans à l'islam des origines, au salaf.

perdus par la République. Nous n'y parviendrons pas en creusant le vide de la France, en désignant la France comme une éternelle coupable, comme un anti-modèle, comme un contre-exemple. Comment voulez-vous agréger ces jeunes générations à la France si vous la présentez comme peu estimable, comme toujours coupable du pire des crimes, celui contre l'humanité ? Monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est grâce à l'épaisseur de notre culture, à la profondeur de notre civilisation et à la hauteur de notre message à la fois singulier et universel que nous parviendrons à agréger ces plus jeunes générations issues de l'immigration à notre destin national. Réaffirmer les principes de la République, oui ; faire aimer la France, c'est plus difficile, mais c'est fondamental

cela a été rappelé, ce texte concrétise le programme de lutte contre les séparatismes dessiné par le Président de la République lors de son discours aux Mureaux. Il porte des avancées importantes, nécessaires et attendues. En introduction aux débats, nous voudrions faire part de notre étonnement sur la motion qui a été déposée et selon laquelle il n'y aurait pas lieu de délibérer. Quelle surprise ... Certaines prises de position de ces derniers jours nous rappellent pourtant qu'il y a urgemment besoin de débat en la matière, de débat auquel toutes les citoyennes et tous les citoyens peuvent participer dans une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Je consacrerai mon court propos au champ éducatif. Nous voterons l'article 1 , qui inclut dans la formation des enseignants et des personnels de l'éducation une formation au principe de laïcité. de laïcité. Nous voterons le renforcement des contrôles sur les établissements d'enseignement privés hors contrat, le renforcement des sanctions à l'encontre des chefs d'établissement d'enseignement privés hors contrat méconnaissant des mises en demeure et la signature d'une charte des valeurs et principes républicains.

Oui, l'autorité déconcentrée doit travailler avec les établissements publics et privés sous contrat d'un même bassin de vie et avec les collectivités territoriales concernées pour améliorer la mixité sociale au sein de ces établissements. Oui, la commission de concertation chargée d'examiner les contrats d'association doit veiller au développement de la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements privés sous contrat. Oui, enfin, au transfert aux conseils départementaux des données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de la circonscription. Faisons toutefois attention, mes chers collègues, de ne pas participer à ce que j'appellerai un effet mikado, c'est-à-dire beaucoup parler pour finalement décevoir. Trop d'attentes ont été déçues ces trente dernières années. Alors que nous tirons continument la sonnette d'alarme sur les effets délétères des inégalités sociales en France et sur le manque de mixité dans les grandes zones urbaines et rurales, en particulier dans nos écoles, faisons preuve non seulement d'un grand volontarisme,

les associations cultuelles qui profitent de ces dispositions extrêmement larges pour proposer des déductions fiscales alléchantes. Beaucoup d'associations passent entre les mailles du filet.

des financements accordés en indiquant que les fonds avaient été transférés directement du compte de l'ambassade vers les entreprises qui ont effectué les travaux de construction sur rapport de l'architecte du projet. Si l'on veut suivre les financements étrangers, c'est assez facile : il suffit de réunir les ambassades étrangères et de leur demander d'appliquer un guide de bonne conduite, comme celui de l'ambassade d'Arabie saoudite ou celui du Koweït.

qui explique que l'État peut parfaitement aider le culte musulman sur plusieurs aspects : « il convient donc d'accompagner la communauté musulmane avec exigence, mais c'est d'abord à elle qu'il revient de s'organiser

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la République est une belle idée, un bel idéal, celui d'une communauté nationale une et indivisible dans laquelle chacun a sa place, quelle que soit son origine, ses moyens, ses talents.

Nous ne sommes pas sûrs que votre projet de loi respecte ces précautions élémentaires. Nous craignons que le texte qui sortira du Sénat n'aggrave encore ce sentiment. Pourtant, plusieurs dispositions vont dans la bonne direction. Je pense à celles qui sont relatives au respect de la laïcité, si essentielle pour nous mais malheureusement trop souvent attaquée, et à celles qui confortent la neutralité du service public. Nous approuvons aussi l'idée de mieux contrôler les financements étrangers des associations cultuelles, ainsi que le fonctionnement des établissements hors contrat. des ambiguïtés subsistent dans votre projet de loi. Nous aurions aimé y trouver des mesures pour renforcer la mixité sociale à l'école, car c'est là que tout commence pour inculquer les principes de la République. Mais, depuis quatre ans, rien n'a été fait dans cette direction, alors que notre école, sur de nombreux plans, est porteuse de ségrégation et de séparatisme. Votre texte reste, hélas ! muet sur ce sujet. Pour nous, l'instruction c'est d'abord à l'école de la République. L'école, c'est le creuset de la République où commence l'apprentissage de la citoyenneté, enrichie par la mixité sociale et le vivre-ensemble. à l'école que commence à se construire la communauté nationale, mais aussi grâce aux activités associatives, pendant les temps périscolaires, et dans les colonies de vacances, trop peu soutenues aujourd'hui pour que les enfants de ce pays apprennent à se connaître, à se respecter et à vivre ensemble. Ce n'est pas la création d'un service national universel, coûteux et inutile, qui résoudra la question de la formation citoyenne des jeunes. Certes, par l'article 21, vous souhaitez resserrer les contraintes sur l'instruction en famille

La droite sénatoriale ayant supprimé cet article 21 en commission, le groupe socialiste va soutenir le Gouvernement. Nous proposerons de rétablir cet article, que nous améliorerons. En contrepartie, nous attendons votre soutien pour enfin légiférer sérieusement sur la création des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat, en exigeant l'autorisation préalable de l'État et du maire avant toute ouverture, par simple cohérence et parallélisme des formes avec votre article 21 originel. Monsieur le ministre, l'engagement associatif sous toutes ses formes est sans aucun doute l'un des piliers les plus authentiques de la démocratie et l'un des exercices les plus aboutis de la citoyenneté. Par l'article 6 de votre projet de loi, vous souhaitez mettre en place un contrat d'engagement républicain, qui reste flou et dont l'utilité est tout à fait discutable. Il nous semble plus opportun de reconnaître dans la loi la « charte des engagements réciproques », qui remplit déjà ce rôle contractuel depuis 2001. Pourquoi voulez-vous encore corseter un monde associatif fragilisé et en souffrance par des contraintes inadaptées et contraires à l'esprit de la loi de 1901 ? Quant à l'article 8, il fait peser de nouvelles responsabilités écrasantes et injustes sur les épaules des dirigeants associatifs, et notamment les jeunes, au motif qu'un comportement inadapté d'un membre pénaliserait l'association tout entière, ainsi que ses dirigeants. Les associations s'en inquiètent. Il me semble que la réglementation actuelle permet déjà d'intervenir.

On y traite de l'héritage, de la polygamie, des mariages forcés, des imams détachés, du droit d'association, des certificats de virginité, des réseaux sociaux, de l'école à la maison, de la liberté du culte et de beaucoup d'autres questions. Je félicite nos rapporteures d'en être venues à bout et d'avoir même réussi à l'enrichir. Beaucoup de mesures parmi celles que le Gouvernement propose méritent d'être retenues. Leur convergence peut donner sens à ce projet de loi, sans qu'il soit nécessaire de lui prêter une portée qu'il ne saurait avoir. L'approche retenue n'est pas gage de lisibilité. De nombreux régimes juridiques vont ainsi être revus à l'aune de la lutte contre l'islamisme radical, en impactant des pratiques profondément ancrées dans notre vie sociale, qui ne sont nullement blâmables et qui, pour certaines d'entre elles, comme celles qui se rattachent à la liberté d'association, ont une valeur civique qui les rend dignes d'être encouragées et non entravées. Ce texte va créer des formalités, des obligations, des contrôles, des restrictions. Il nous est demandé de faire accepter aux Français le sacrifice d'une part de liberté au nom du combat, salutaire, contre l'islamisme radical. Cela ne peut se faire de gaieté de coeur, même si la cause est juste. Pour en arriver là, le Gouvernement invoque un argument qui ressemble à une excuse à cause du principe d'égalité, on ne peut faire une loi sur l'islam et ses associations. Il faudrait donc, selon lui, faire une loi sur tous les cultes et sur toutes les associations. Cette approche me paraît contestable. Nous n'avons pas plus besoin d'une loi sur l'islam que d'une loi sur la religion en général pour faire reculer l'islamisme : ce combat est en effet un combat politique ... Tout Ce que nous appelons police des cultes n'est pas une police des croyances- elles sont libres ! -, c'est la police de la séparation du politique et du religieux voulue par la loi de 1905, dont les principes et les règles demeurent d'actualité. Toute assimilation entre chrétiens d'hier et islamistes d'aujourd'hui serait historiquement fausse, chère Dominique Vérien. Ce que la République doit viser, ce sont les dérives dogmatiques d'un segment dévoyé de l'islam qui conteste nos lois et notre Constitution. Il s'agit de menées idéologiques. Nous avons voulu, au Sénat, les tenir en échec par la reconnaissance d'un nouveau principe constitutionnel applicable à l'ensemble des situations dans lesquelles les salafistes avancent leurs pions : à l'école, à l'hôpital, dans les centres sportifs et culturels et les associations, sur les lieux de travail, dans la vie en société Vous ne l'avez pas voulu. Vous avez eu tort ; nous n'y avons pas renoncé. S'agissant des cultes, nous avons déjà des moyens d'action importants, qu'il n'est pas interdit de consolider : fermeture de mosquées, expulsion d'imams étrangers, condamnation des incitations à la haine, pénalisation de toute mise en cause de la loi par un ministre du culte ... Tout ce qui va dans ce sens peut aisément être approuvé. Toutefois, au cours des dernières années, le Gouvernement ne semble pas avoir essayé de mettre en oeuvre les sanctions de la loi de 1905, qui permettent de punir l'intrusion d'imams dans le champ politique point de volonté gouvernementale, point de consignes aux préfets ni aux procureurs. La justice n'est jamais saisie. La loi paraît oubliée de ceux-là mêmes qui sont en charge de l'appliquer : sans volonté politique, à quoi servirait-il de la changer ? Le Sénat a, de longue date, sonné l'alarme devant les progrès du salafisme, qui portent atteinte à l'unité de la Nation. Toute complaisance à son égard relève d'une forme de complicité. Ce projet de loi risque pourtant de n'être qu'un tigre de papier, car on n'arrête pas les idéologies par des barrières bureaucratiques ou budgétaires. Les valeureux agents de nos préfectures et de nos directions des finances publiques dépouilleront avec un soin méticuleux les déclarations des cultes. Mais quoi de plus facile que de respecter les formes et les déclarations d'intention qu'exigent les articles les plus naïfs de ce texte ? Il y aura plus de contraintes pour ceux qui inscriront leur action dans le cadre légal et plus d'hypocrisie ou de clandestinité pour les autres. Régir les lieux de culte et leurs abords est une chose, mais le champ d'action des islamistes radicaux ne s'arrête pas là : il s'étend à la rue, aux associations, aux réseaux sociaux et aux lieux d'habitation. Pour tout dire, monsieur le ministre, je ne crois pas à l'efficacité globale de votre texte. J'admets qu'il marque une certaine prise de conscience de la gravité des forces centrifuges qui menacent notre nation. Il constitue, à ce titre, un tournant dans la politique du Gouvernement. Le Président de la République paraît être enfin passé de l'éloge du multiculturalisme à une vision plus exacte des menaces qui pèsent sur le vivre-ensemble. C'est un premier pas. Malgré les défauts de conception de ce projet de loi, nous pourrions vous laisser votre chance si vous acceptiez nos principaux amendements.

Premier principe : la liberté de culte. Elle est totale en France. La laïcité garantit la liberté d'exercice des cultes.

articles de ce projet de loi, l'État, d'une certaine manière, organise les cultes. Troisième principe : l'État fait respecter la loi de la République.

en accroissant les contraintes sur la loi de 1905, vous ferez que ceux qui sont régis par la loi de 1901 désirent s'inscrire dans ce cadre ? Pour ma part, je n'en suis pas du tout sûr.

Parce que, tout le monde en est conscient, à force de coups de canif, à force de coups de poignard, les Français se demandent s'il y a encore une République dans ce pays,

l'accumulation et la force de ces coups de canif contre la République qui remettent en cause l'adhésion à la République et la force de la République. Or si la République ne doit être ni de gauche ni de droite, elle doit être respectée par tous. Monsieur le ministre,

Incontestée, cela ne veut pas dire que tout le monde doit avoir la même opinion, la même religion ou la même organisation. Notre pays a toujours connu- heureusement ! -des débats démocratiques

des coups de canif remet gravement en cause la stabilité de la République et sa durée. Que personne ne s'illusionne, aucun régime politique

Oui, c'est un fait, les tentations séparatistes pénètrent la République en son coeur le plus sacré, l'école, laquelle constitue de moins en moins l'asile inviolable espéré par Jean Zay ! Oui, c'est un fait, les tentations séparatistes menacent l'éducation de la jeunesse de France bien entendu à l'existence d'enfants « hors radars » de l'obligation d'instruction, qui ne sont ni ceux de l'école publique ou privée ni ceux de l'instruction en famille, lesquels sont parfaitement connus, identifiés, déclarés et recensés. bien aux écoles de fait, ces établissements clandestins qui se développent, sans même avoir besoin d'utiliser le faux nez de l'instruction en famille. Je pense aussi aux pressions auxquelles sont confrontés enseignants et chefs d'établissement au coeur même de l'école publique, où l'islamisme déstabilise les professeurs et les enseignements, la vie scolaire et la vie périscolaire et même le vivre-ensemble entre les garçons et les filles.

Or, dès le 15 janvier 1850, Victor Hugo, déclarait : « À côté de cette magnifique instruction gratuite, [ ...], je placerais sans hésiter la liberté d'enseignement, la liberté d'enseignement pour les instituteurs privés, la liberté d'enseignement pour les corporations religieuses ; la liberté d'enseignement pleine, entière, absolue, soumise aux lois générales comme toutes les autres libertés, et je n'aurais pas besoin de lui donner le pouvoir inquiet de l'État pour surveillant, parce que je lui donnerais l'enseignement gratuit de l'État pour contrepoids.

Alors même que vous avez été incapable, au-delà des cas d'espèce, d'étayer le moindre corollaire entre instruction en famille et menaces séparatistes,

les parents sont présumés coupables de ne pas poursuivre l'intérêt supérieur de leurs propres enfants, et la puissance publique est jugée seule apte à le définir. Nous passons bien d'un contrôle que je ne discute pas, un contrôle sociétal de l'intention et de la motivation même des parents. Aussi notre commission a-t-elle eu la sagesse de supprimer l'article 21, tout en introduisant un certain nombre d'éléments permettant de renforcer les contrôles en cas de doute sérieux. Notre commission a ainsi rappelé avec force que la liberté de choix des parents ne peut être aliénée. Elle Elle a aussi rappelé avec force que les parents sont les premiers et les ultimes éducateurs de leurs enfants. Elle a surtout rappelé que la coexistence de propositions éducatives variées est le signe d'une société démocratique plurielle, respectueuse de la diversité, laquelle n'exclut pas la concorde nationale. Mes chers collègues, à rebours du « pouvoir inquiet de l'État », je souhaite que l'examen de ce texte soit l'occasion de changer de paradigme pour mieux contrôler ce qui doit l'être, sans faire peser sur les familles qui ne font pas le choix de l'école publique une insupportable présomption de culpabilité. Si nous devons mieux armer l'école publique et ses « hussards noirs », en améliorant leur formation ou en rompant avec la culture du « pas de vagues », si nous devons nous mobiliser pour que l'instruction publique demeure un contrepoids et redevienne porteuse de promesses et d'avenir pour les enfants de ce pays, ce n'est pas en se reniant et en se que la République luttera contre le séparatisme. Car s'il devait y avoir, comme le proclamait Clemenceau, un conflit entre la République et la liberté, c'est bien la République qui aurait tort. Très bien ! Très belle citation ! C'est au contraire en réaffirmant son attachement viscéral à nos libertés fondamentales et, parmi elles, à la liberté d'enseignement « pleine, entière, absolue, soumise aux lois générales comme toutes les autres libertés », que la République puisera sa plus haute force.

J'ai découvert, quand j'étais maire- je suis sûr que c'est arrivé à chacune et chacun d'entre vous dans les territoires les plus compliqués -, des petits fantômes de la République. En 2019, sur les 50 000 enfants qui étaient instruits en famille, 25 000 l'étaient pour des raisons médicales.

se posent naturellement des questions ; ils se demandent s'ils sont les bienvenus dans la République, si l'on respecte la vie de leurs parents et de leurs grands-parents et si leurs enfants pourront vivre de manière

le communautarisme, en particulier le communautarisme religieux- mais pas seulement -, sur les principes de la République. Tout ce qui est contenu dans ce texte cible ouvertement ou implicitement les séquelles du communautarisme. Il faut appeler un chat un chat ! Or on a peur de dire que, si nous sommes tous réunis ici,

face au communautarisme, qu'il soit religieux ou autre, car là est le vrai problème qui se pose actuellement.

de leurs milieux sociaux. Nous avons concentré les difficultés économiques et éducatives dans certains quartiers de la République. Nous avons ainsi créé des quartiers où la promesse de République n'a pas été tenue. reflète le fait que la société n'a pas apporté le minimum nécessaire à tout un pan de la population. La casse du service public, le chômage massif, la précarité et la pauvreté se et montrent justement que les devoirs minimaux d'un pays riche comme la France, envers son peuple, ont été négligés. Pour toutes ces raisons, nous demandons que cet amendement soit adopté. Quel est l'avis de la commission ? La notion

le 12 avril 1905, disait : « Par la deuxième partie de l'article 1, la République, envisageant les manifestations extérieures des croyances et des religions, qui constituent l'exercice des cultes, s'engage à en garantir la pleine et entière liberté. » La liberté de culte s'entendait alors comme la faculté pour chaque individu de pratiquer sa croyance ou, en d'autres termes, d'exercer par des actes extérieurs le culte qu'il a choisi.

et liberté de culte. Mon parcours personnel ainsi que la famille et la tradition politiques auxquelles j'appartiens me font croire que la spiritualité est indissociable de ce qui a fait la France, par sa culture et l'histoire de ses idées. Par conséquent, je remercie Nathalie Goulet d'avoir déposé cet amendement,

qui protège celle de croire ou de ne pas croire, sans la menace de se voir imposer d'autres convictions. La République assure la liberté de conscience, et l'État, par sa neutralité, en se tenant en dehors du champ des options spirituelles et confessionnelles,

extérioriser, d'une manière ou d'une autre, une sympathie ou une antipathie quelconque, comme on le voit trop souvent ! Quel est l'avis de la commission ?

Dans le même temps, vous avez indiqué que le maire était à la fois agent de l'État et élu de la collectivité. Lorsqu'un maire célèbre un mariage, il officie en tant qu'agent de l'État.

à ce qui fait l'essence du droit local, c'est-à-dire les dispositions existantes applicables aux cultes reconnus.

le culte catholique, les deux cultes protestants, calviniste et luthérien, et le culte israélite -et des cultes non reconnus, dont le culte musulman, mais pas uniquement. Nous

Si vous ne faites pas la différence entre les musulmans et les islamistes, c'est que vous avez un gros problème. Moi, je n'ai pas ce problème ! Je suis fier de stigmatiser les islamistes, de viser ceux qui arment les esprits des terroristes. Alors, disons-le : oui, nous devons nous attaquer aux islamistes ! Pour ne pas stigmatiser les cultes, il faut désigner l'ennemi. En refusant de le nommer, vous vous attaquez aussi aux cultes catholique, protestant ou juif, qui sont très inquiets de votre texte. Avec cet amendement, je vous propose de désigner l'islamisme de manière très précise, sur le fondement de critères objectifs, clairs et totalement légaux. L'islamisme se caractérise par son mépris de nos lois et de la dignité humaine. Il refuse toute liberté de conscience ou d'expression, combat notre démocratie, soutient clairement, ou à demi-mot, les actes terroristes, les appels à la haine contre les non-croyants. L'islamisme existe, et le Président de la République est allé plus loin en évoquant précisément les courants salafistes, wahhabites ou issus des Frères musulmans, qui sont les plus virulents dans notre pays. On pourrait évidemment y ajouter l'association Millî Görüs, proche du dictateur Erdogan, qui fait construire une mosquée géante à Strasbourg, mosquée que la mairie islamo-écolo veut subventionner et dont le chantier avait été inauguré par la députée européenne Les Républicains Fabienne Keller. Vous le voyez, il ne faut pas avoir peur des mots ; il faut dire les choses, nommer les responsables et les coupables, les complices, sans oublier, bien sûr, les idiots utiles. Si le Président de la République peut le dire, pourquoi avons-nous, nous, peur de le faire ?

que vous faites partie de ces personnes. Cet amendement évoque par ailleurs « l'incompatibilité radicale qui peut exister entre ces idéologies et les droits, libertés et principes reconnus ou consacrés par la Constitution, et notamment la dignité humaine ». Vous devez être ravi, monsieur le ministre : c'est là le meilleur argument pour justifier la dissolution de Génération identitaire

projet de loi. Le discours prononcé aux Mureaux en octobre dernier par le Président de la République était fort, les mots sonnaient juste. À dix-huit mois de la fin de son mandat, le Président de la République semblait avoir pris la mesure du danger mortel qui menace notre nation. Mais, alors que le projet de loi confortant les principes de la République est examiné par le Parlement, que reste-t-il du discours des Mureaux ? Peu de choses ... La dénonciation de l'islamisme a pudiquement laissé place à celle du séparatisme, puis à la défense des principes républicains. Alors que notre ennemi, c'est le totalitarisme islamique,

Philippe Bas. L'État aura un droit de regard sur les agissements des associations et sur leur financement. Oui, la polygamie et les certificats de virginité feront l'objet d'une vigilance particulière. Oui, les agents administratifs et les enseignants seront davantage protégés. Mais, quand on veut lutter contre le totalitarisme islamique, il faut légiférer sur l'immigration, exiger plus d'assimilation et réaffirmer haut et fort notre conception humaniste et universaliste du monde. Le mot « universalisme » me semble essentiel.

L'actualité nous oblige à parler de ce qui se passe aujourd'hui à Strasbourg. Alors que nous assistons, dans une capitale européenne, à la construction de la plus grande mosquée d'Europe, commanditée, ou en tout cas très soutenue

: le principe de liberté, mais aussi le principe d'égalité et le principe de fraternité. Lorsque l'un des piliers de notre devise républicaine s'effrite, c'est l'ensemble de la République qui s'affaiblit. C'est, hélas ! l'une des choses que nous observons aujourd'hui : l'égalité recule, la République avec elle. Cela fait des années que les inégalités sociales s'accroissent dans notre pays et que la promesse républicaine s'érode, en particulier dans la jeunesse.

aucun arsenal législatif pour les accompagner dans la gestion des relations avec les représentants religieux et mettre fin à toute forme d'accommodement local. Or nos élus locaux sont les premiers dépositaires des principes fondateurs de notre République et sont en première ligne pour leur mise en oeuvre. La laïcité transparaît derrière chacune de leur action. Toutefois, comme j'ai pu le constater dans mon département lors de mes déplacements en mairie, en matière de laïcité, il y a la théorie et la pratique, l'application stricte des textes et la voie tracée par la jurisprudence. Les deux doivent être appréhendés concomitamment. La sensibilisation et la formation de nos élus sont donc indispensables. Pour ma part, j'ai rédigé un petit guide pratique de la laïcité à destination des 535 maires de la Gironde, de leurs équipes municipales et de leurs agents afin de leur donner les outils nécessaires pour appliquer ce principe, que ce soit pour les prêts de salles, la gestion des lieux de sépulture

aux agents titulaires de la fonction publique et des services publics, mais aussi à tous ceux qui participent au service public. Il est réellement intolérable

Néanmoins, si la question du port de signes religieux lors des sorties scolaires fait souvent débat, il n'est pas nécessaire de fixer exclusivement notre attention sur ce point très spécifique. En effet, cette problématique touche l'ensemble de la catégorie juridique des collaborateurs occasionnels du service public, catégorie dont le statut a été largement déterminé par la jurisprudence du Conseil d'État. Aussi, puisque la neutralité du service public est un principe essentiel devant être défendu, il est nécessaire qu'elle s'applique à toute forme de mission, indépendamment du statut juridique de celui qui l'exerce. L'objet de cet amendement est d'étendre au-delà des seuls fonctionnaires, agents contractuels ou extracontractuels, l'obligation de s'abstenir de manifester ses opinions politiques ou religieuses, de traiter de façon égale toutes les personnes et de respecter leur liberté de conscience et leur dignité. L'amendement n° 60 rectifié,

aux agents, mais également aux usagers. Il faut poursuivre dans cette longue et belle histoire de l'école laïque. Une sortie scolaire est un acte pédagogique ; c'est l'école hors des murs. Ceux qui participent à cet acte pédagogique en aidant les professeurs et en accompagnant les élèves doivent donc afficher une stricte neutralité politique, philosophique

c'est un bien petit sacrifice face à un grand principe. Voilà pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement, qui vise à renforcer la neutralité politique et religieuse de notre école, dans et hors ses murs. L'amendement

Pour une fois, j'irai dans votre sens. Oui, Nicolas Sarkozy a raison : personne ne comprend que le voile islamique soit autorisé à l'université ! Alors, agissons agissons sans avoir peur et interdisons-le ! Dans le temple du savoir et de la connaissance qu'est l'université, on ne saurait tolérer un tel symbole d'asservissement de la femme. Les femmes se sont battues pendant des siècles pour leur liberté. Ayons le courage de la protéger à l'heure où les islamistes la remettent en cause Accepter le voile à l'université, c'est laisser le champ libre aux revendications islamiques de tous ordres ; c'est la première reculade avant la capitulation ! Je ne suis d'ailleurs pas le premier à réclamer une telle interdiction ; le Haut Conseil à l'intégration l'avait La laïcité ne se divise pas. Elle se vit entièrement, pleinement, d'un bloc. Il n'y a pas une laïcité pour l'école et une laïcité pour l'université. Il n'y en a qu'une seule celle de la République ! Chers collègues de gauche, soyez fermes face à l'islamisme ! Je sais que la mode chez vous est à la compromission et au relativisme. Mais l'enjeu est trop grand. Ne faites pas une fois de plus reculer la République Tout accepter, c'est concéder la victoire à nos ennemis, c'est-à-dire les islamistes ! Si vous tolérez aujourd'hui le voile à l'université, pourquoi ne pas accepter demain les cours séparés pour les femmes voilées ? Chers collègues de droite, soyez cohérents ! J'ai l'habitude de défendre des textes que vous réclamez, mais que vous n'osez pas assumer.

À l'heure où une récente enquête de l'IFOP pour la Licra révèle une jeunesse majoritairement favorable à l'expression de la religiosité en public, considérant ainsi la laïcité comme une forme de discrimination envers les musulmans, le Parlement doit se prononcer sur le cas des parents participant aux sorties scolaires de leurs enfants. Le renforcement de la neutralité du service public étant l'un des objectifs du présent projet de loi, l'occasion nous est ainsi offerte de pouvoir décliner cette neutralité dans le cadre des sorties et activités scolaires. Actuellement, le code de l'éducation dispose que, dans les établissements scolaires, la manifestation ostensible d'une appartenance religieuse par les élèves est interdite, qu'il s'agisse de signes ou de tenues. Néanmoins, la situation des parents accompagnateurs dans les sorties scolaires est ignorée. Or, dans la mesure où le parent d'élève reçoit au cours d'une sortie scolaire une délégation d'autorité de l'enseignant sur les enfants, le principe de neutralité religieuse qui s'impose à l'enseignant doit être étendu à l'ensemble des activités réalisées pendant le temps scolaire lorsqu'elles sont assurées par le parent d'élève. En tant que collaborateur occasionnel du service public, le parent d'élève devrait se voir transposer les obligations du service public : toute manifestation d'appartenance religieuse devrait donc lui être interdite. À ce sujet, je regrette que l'avis des rapporteures n'ait pas été entendu

la laïcité française, qui n'est pas la neutralité dans l'espace public. Exactement ! La laïcité française est au contraire l'acceptation de la pluralité religieuse et des expressions, même religieuses, y compris si elles nous embêtent.

Mme la rapporteure.

l'amendement que M. Brisson souhaite faire voter ne pourrait pas, me semble-t-il, résoudre le problème. En l'espèce, le Conseil d'État pourrait prendre exactement la même décision

les personnes qui accompagnent les enfants dans les sorties scolaires ou, éventuellement, qui entrent dans l'école sans exercer de mission d'enseignement ne sont pas soumises au principe de neutralité. À ce titre, elles peuvent, comme dans l'espace public en effet, arborer des signes d'appartenance à telle ou telle religion dès lors qu'elles s'abstiennent de faire du prosélytisme.

Comme le souligne Kahina Bahloul, imam, femme et non voilée, dans un livre que je vous invite à lire, le voile ne relève pas d'une obligation religieuse. C'est une tradition issue de l'interprétation des textes qui, certes- nous en convenons et nous le condamnons -, est une marque de soumission de la femme. Mais, pour l'immense majorité d'entre elles, cas un acte politique. Mes chers collègues, je préfère une maman qui marche avec la République en accompagnant son enfant à l'école laïque aux familles qui, se sentant stigmatisées, mettraient leur enfant dans une école confessionnelle ou préféraient l'instruction en famille, celle-là même que vous allez rétablir tout à l'heure. Attention à ne pas pointer du doigt l'immense majorité silencieuse de nos compatriotes musulmans, qui vivent leur religion de façon paisible et sans faire de bruit ! Au-delà, faudra-t-il appliquer le principe de laïcité

déclinés sur plusieurs modes : les accompagnatrices scolaires, les piscines ou encore les assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Le positionnement qu'ils impliquent ne saurait être dogmatique, mais pourrait s'articuler autour de deux questions dont nous pourrons, me semble-t-il, assez largement partager la nécessité. Premièrement, y a-t-il un vide juridique à combler ? Il semble que le Conseil d'État ait apporté des éléments éclairants dans son avis de 2013, lorsqu'il a déclaré que « les exigences liées au bon fonctionnement de l'éducation peuvent conduire l'autorité compétente, s'agissant des parents d'élèves qui participent à des déplacements ou des activités scolaires, à recommander de s'abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses ». La manifestation des convictions religieuses a pour limite le trouble à l'ordre public, comme le précisait M. le ministre, ou le bon fonctionnement du service public. Faut-il substituer à ce critère, qui implique un discernement casuistique, une interdiction générale et absolue ? Je ne le pense pas.

Permettrait-elle de faire obstacle à la pression interne à la société française visant à fermer une partie de la société aux valeurs de la République ? Je ne le pense pas non plus. La laïcité, dont est déduite la liberté de conscience, n'est pas le silence des opinions religieuses des personnes appréhendées comme usagers du service public. Il ne s'agit pas ici de mollesse ou de renoncement, mais de porter une interrogation simple au regard de l'objet du texte. Il s'agit aussi que le principe de laïcité ne doit pas nécessairement sentir la poudre, pour reprendre les mots de Jean Rivero, mais peut constituer un principe fédérateur rassemblant l'ensemble des citoyens, croyants ou incroyants, comme l'exprimait Jean-Marc Sauvé. Ne manquons pas notre cible, mes chers collègues ! Pour ces raisons, vous l'aurez compris, le groupe RDPI ne votera pas ces amendements.

lorsque nous aborderons les amendements visant à rétablir l'article 21. En revanche, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas parlé de collaborateurs occasionnels ni de signes ostentatoires ou ostensibles.

dans un espace de découverte, ils apprennent aussi la laïcité. Comme l'a dit M. Badinter, pour les mamans ou les papas qui participent à cet acte pédagogique, ce n'est pas un grand sacrifice

! Ils n'entrent pas dans l'école- ou hors l'école -seulement à l'occasion des sorties scolaires. Les mères que vous visez en vérité à travers ces amendements sont extrêmement présentes dans l'éducation de leurs enfants et dans l'école publique.

Je ne le crois pas. Il y a selon moi des combats plus importants à mener à l'encontre de l'islamisme radical.

de l'autre. Ce n'est pas un hasard si, au cours des trois derniers quinquennats- le second mandat de Jacques Chirac avec la loi de 2004, le quinquennat de Nicolas Sarkozy avec la loi de 2010, celui de

y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l'enseignement dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles et établissements publics locaux d'enseignement ». Il ne s'agit donc pas des parents d'élèves ou des intervenants qui viennent collaborer de temps en temps, mais des personnes qui « participent

mes chers collègues. Monsieur Brisson, comment pouvez-vous dire que les accompagnatrices ou les accompagnateurs de sorties scolaires exercent directement une mission de service public ? Ils ne

initiateur de cette loi, assurait que l'État n'avait pas à se soucier de la signification religieuse d'un vêtement.

laïcité. La laïcité, c'est aussi la tolérance vis-à-vis de l'ensemble des cultes, quand bien même ils me gêneraient en tant qu'athée, agnostique ou membre d'une autre croyance.

dans l'école laïque en accompagnant son enfant. Si vous privez ce parent de cet accompagnement, vous privez non seulement l'enfant, mais vous risquez également de priver toute la classe, car les parents accompagnateurs ne sont pas pléthoriques. Vous commettez vraiment, me semble-t-il, une faute grave.

vocation à irradier toute la société française. La République est laïque ; la société et les individus ne le sont pas. Les parents sont très souvent sollicités

que ce soit avec des arrière-pensées prosélytes, mais tout simplement pour rendre service. Je voudrais lever deux ambiguïtés qui ont pu naître de nos échanges. Premièrement, ces accompagnatrices ne participent ni à l'enseignement

des enseignants et des directeurs qui organisent les sorties scolaires. Or il serait utile de savoir quelle est leur position et nous sommes assez nombreux à avoir

Monsieur le ministre, dans votre long exposé en appui de l'avis que vous avez donné sur ces amendements, vous avez recouru à une surabondance d'arguments, ce qui, de mon point de vue, affaiblit votre raisonnement. Quand on a un raisonnement fort, on n'a pas besoin de rajouter des arguments aux arguments. Premièrement, ces amendements concernent l'école publique. Vous leur reprochez de ne pas concerner l'école privée, mais il d'une donnée fondamentale de la liberté de l'enseignement : le caractère propre des établissements privés fait que nous ne devons pas leur appliquer les mêmes règles qu'aux établissements publics, ou alors il faut remettre en cause la liberté de l'enseignement. Deuxièmement, la distinction entre l'activité pédagogique hors les murs et celle dans les murs ne tient pas debout. Le professeur est neutre dans les murs, il l'est aussi hors les murs ! Parce qu'il est professeur ! Et il n'y a pas d'obstacle à ce que, si nous le décidons, l'accompagnateur de sortie scolaire se voie imposer des obligations de neutralité quand il participe avec le professeur à des activités pédagogiques hors les murs. Troisièmement, ces parents, contrairement à ce que j'ai entendu, ne sont pas des usagers du service public. Ils ont une mission : ils ne se bornent pas à s'occuper de leurs propres enfants, ils s'occupent aussi des enfants des autres ; ils exercent,

respecter la liberté de l'enfant, en évitant de l'exposer à une forme d'influence psychologique exercée par une certaine revendication d'appartenance religieuse qui s'imposerait

Par conséquent, je crois que les arguments qui nous sont opposés n'ont que peu de consistance

religieuse : « L'emploi, par diverses sources et pour des finalités diverses, de la notion de " collaborateur ", de " collaborateur occasionnel " ou de " participant " ne dessine pas une catégorie juridique, dont les membres seraient, entre autres, soumis au principe de neutralité religieuse. »

je lui dirai que le silence du projet de loi au sujet du costume ecclésiastique, qui paraît le préoccuper si fort, n'a pas été le résultat d'une omission, mais bien au contraire d'une délibération mûrement réfléchie.

que de vouloir, par une loi qui se donne pour but d'instaurer dans ce pays un régime de liberté au point de vue confessionnel, d'imposer aux ministres des cultes l'obligation de modifier la coupe de leurs vêtements. Je ferai du reste observer à l'honorable M. Chabert que le problème n'est pas aussi simple ni aussi facile à résoudre qu'il semble le supposer. Ce que notre collègue voudrait atteindre dans la soutane, c'est le moyen qu'elle procure de se distinguer facilement des autres citoyens. » On pourrait évidemment reprendre cet argument pour celles qui se distinguent par le voile islamique, Mais la soutane une fois supprimée, M. Chabert peut être sûr que, si l'église devait y trouver son intérêt, l'ingéniosité combinée des prêtres

Alors, c'est sciemment que j'ai refusé ces dispositions, considérant que la loi d'interdiction de l'intolérance, mais d'autorisation de la liberté, permettait au Parlement d'assouvir ce que la République voulait.

celui du Gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.